La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 9 novembre 2017 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation

En 1947, Jack Ralite adhère au parti communiste français. Épris de littérature dès l'adolescence, il intègre la rédaction de dont il dont il devient plus tard responsable des pages culture, presque naturellement. En 1959, notre ancien collègue est élu au conseil municipal d'Aubervilliers, il sera maire pendant près de vingt ans, de 1984 à 2003. Député de la Seine-Saint-Denis de 1973 à 1981,

et devient l'un des piliers de la commission de la culture. La culture, qu'il considère comme un outil d'émancipation, est en effet le fil rouge de son engagement politique. À Aubervilliers, il est à l'origine de la création, dès 1960, du théâtre de la Commune, premier centre dramatique de la petite couronne. Au sein de notre hémicycle, sa mobilisation aura été constante pour défendre artistes, éducation, accès à la culture, exception culturelle ou encore télévision de qualité. Ceux qui l'ont connu comme moi au sein de notre assemblée se souviennent d'une grande voix, d'une forte voix, d'une expression toujours chaleureuse, d'un homme de conviction et au goût marqué pour les citations. Dans l'un de ses discours, il avait ainsi cité Pierre Boulez

Cette phrase s'applique parfaitement à Jack Ralite. Au nom du Sénat, je veux présenter nos condoléances les plus attristées à sa famille et assurer ses proches, la présidente et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste,

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2018

le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale de cette mandature. Ce PLFSS est à la fois un texte dense et un texte qui fait des choix. fait le choix du pouvoir d'achat pour les salariés par la baisse des cotisations sociales et par l'augmentation, au 1 octobre prochain, de la prime d'activité. fait le choix de conforter notre modèle de protection sociale en adaptant son financement à l'évolution de notre économie et de notre société et en renforçant son universalité, afin que chacun puisse bénéficier de la même sécurité sociale quel que soit son statut professionnel. fait le choix- j'y reviendrai -de la solidarité au bénéfice de nos concitoyens les plus fragiles, qu'il s'agisse des bénéficiaires du minimum vieillesse ou des familles les plus pauvres. Choisir, c'est aussi assumer une politique de prévention ambitieuse qui protège nos concitoyens et prend à bras-le-corps la première des inégalités en matière de santé : l'inégalité devant la prévention. Faire des choix, c'est également poser, dès maintenant, les jalons pour une transformation continue et résolue des modalités de tarification des actes et des prestations qui incitent à privilégier la pertinence et la qualité et qui prennent en compte les besoins des patients dans leur globalité. Les choix que ce PLFSS vous propose sont ceux d'une France qui porte haut l'ambition d'un modèle de protection sociale et d'un modèle de santé solidaires, d'un modèle qui permette l'égal accès aux soins et à l'innovation pour tous, qui garantisse aux citoyens l'équité devant la retraite et qui réponde efficacement aux besoins prioritaires des familles. Ces choix ne sont possibles, ces choix ne sont crédibles, mesdames, messieurs les sénateurs, que si nous nous donnons les moyens de rétablir l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. Je sais votre assemblée très attentive à cet objectif. En tant que ministre des solidarités, je suis particulièrement attachée à ce que nos concitoyens puissent avoir durablement confiance dans leur système de protection sociale. sans équilibre des comptes, il n'y a pas de confiance possible à moyen et à long terme. L'année 2017 verra les comptes de la sécurité sociale s'améliorer de 2,6 milliards d'euros par rapport à 2016, avec toutefois un déficit encore important de 5,2 milliards d'euros. En 2018, le déficit devrait à nouveau se réduire de 3 milliards d'euros par rapport à 2017. C'est une trajectoire en ligne avec l'objectif fixé par le Premier ministre dans son discours de politique générale d'un retour à l'équilibre à l'horizon de 2020. Suivre ce chemin exigeant, c'est certes faire des choix, mais c'est aussi ouvrir à nos concitoyens la perspective nouvelle de la fin du déficit de la sécurité sociale et offrir aux jeunes générations une protection sociale débarrassée de la dette sociale accumulée au cours des vingt dernières années.

Ma première préoccupation concerne les personnes âgées les plus pauvres. Elles sont plus d'un demi-million en France à vivre avec 800 euros par mois. Nous augmenterons donc le minimum vieillesse de 100 euros par mois, conformément aux engagements du Président de la République. Cela commencera dès le 1 avril prochain, avec une augmentation de 30 euros ; l'augmentation sera ensuite de 35 euros en janvier 2019 et de 35 euros supplémentaires en janvier 2020. À mi-mandat, le minimum vieillesse aura donc augmenté de plus de 12 %.

100 millions d'euros seront consacrés au renforcement de l'encadrement soignant. Par ailleurs, j'ai souhaité soutenir, avec ce PLFSS, le déploiement progressif d'astreintes infirmières la nuit. Ce dispositif permet un meilleur traitement des problèmes qui peuvent survenir la nuit et évite ainsi des hospitalisations inutiles dont on sait qu'elles sont toujours très délétères pour des personnes dépendantes et fragiles. Ce PLFSS s'adresse aussi aux familles. Je veux mettre en adéquation les priorités et les outils de la politique familiale avec les besoins des familles. Notre pays se distingue de longue date par l'importance qu'il attache à une politique familiale large et structurée. Cette politique affiche des réussites manifestes : un taux de fécondité parmi les plus élevés d'Europe, une participation relativement forte des femmes au marché du travail et une conciliation entre vie familiale et vie professionnelle qui doit encore progresser, mais qui est facilitée par une offre d'accueil du jeune enfant substantielle, diverse et financièrement accessible. Mais je fais aussi le constat que la politique familiale est aujourd'hui en perte de repères quant à ses finalités et ses priorités, et que le nombre de naissance est en baisse depuis plusieurs années. La politique familiale est un élément essentiel pour faire société et construire le monde de demain. Elle mérite que nous ayons un débat ouvert, large, sur la façon dont elle répond aujourd'hui, concrètement, aux attentes des familles comment augmenter et améliorer les solutions de garde des jeunes enfants et prendre mieux en compte les besoins des parents qui travaillent ou recherchent un emploi ? Comment aider les familles en difficulté éducative et être plus efficace dans le soutien à la parentalité ? Comment contribuer à réduire les situations de pauvreté ? La France compte aujourd'hui trois millions d'enfants vivant dans un foyer dont les revenus se situent en dessous du seuil de pauvreté. Cette réalité, nous devons nous en saisir pour la faire évoluer, et c'est pour moi une priorité. Ce premier PLFSS fait un choix très clair, celui d'augmenter les prestations à destination des familles les plus fragiles. Les familles nombreuses les plus pauvres bénéficieront de la hausse du complément familial majoré au 1 avril 2018- 450 000 familles Pour les familles monoparentales, qui sont souvent parmi les plus en difficulté, le montant de l'allocation de soutien familial sera revalorisé, au 1avril également- 750 000 familles en bénéficieront. Le montant maximal de l'aide à la garde d'enfants pour les parents qui recourent à un assistant maternel, à une garde à domicile ou à une microcrèche, augmentera de 30 %. Ce PLFSS fait des choix, dont certains peuvent faire débat, mais il s'inscrit résolument dans la perspective plus large d'une concertation menée en 2018 avec l'ensemble des parties prenantes, avec les organisations familiales, avec les parlementaires également, pour redéfinir les objectifs assignés à notre politique familiale. Ce PLFSS, je l'ai indiqué, est aussi un PLFSS de transformation : il engage des évolutions structurelles pour les années à venir.

Cette réforme part du constat, largement partagé, que le lien de confiance entre les indépendants et leur régime de sécurité sociale a été durablement altéré par les difficultés de mise en place de l'interlocuteur social unique depuis 2008. Cette réforme s'inscrit aussi dans la perspective d'une sécurité sociale universelle, qui vise à simplifier les démarches des citoyens, quel que soit leur parcours professionnel- salarié ou travailleur indépendant -ou leur statut- je pense notamment aux étudiants. Elle est donc une nouvelle étape de la construction de notre système de protection sociale et une forme de retour aux sources de l'ambition des fondateurs de la sécurité sociale en 1945. Je vous sais légitimement très attentifs aux conditions de mise en oeuvre de la réforme. Parce que c'est une réforme ambitieuse, nous donnons le temps et les moyens nécessaires à la transformation. Vous le savez, au 1 janvier 2018, une période de transition de deux ans sera ouverte. Cette période permettra de faire évoluer progressivement les organisations de travail et de mener un dialogue social de qualité avec les salariés et leurs représentants. Je veux redire devant vous mon attention à l'accompagnement social et professionnel des salariés du RSI, comme de ceux des organismes conventionnés qui servent les prestations d'assurance maladie. Cette période de transition est nécessaire, elle sera même un peu plus longue pour la reprise de l'activité des organismes conventionnés qui n'interviendra qu'en 2020. Elle ne doit pas être prolongée au-delà, de façon à donner aux organisations et aux personnels un cadre pérenne de travail. Elle n'impose pas de date butoir s'agissant de l'évolution des systèmes d'information. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que l'organisation mise en place permette une évolution graduée et maîtrisée de ces systèmes, dans des conditions de sécurité garanties. Je veux enfin dire l'attachement du Gouvernement à la reconnaissance, au sein du régime général, de la spécificité de la situation des travailleurs indépendants, de façon à adapter le service qui leur est rendu.

Elle redonnera de la lisibilité à un système qui s'est construit par strates successives et qui est aujourd'hui devenu complexe et opaque pour les Français. Elle devra également assurer la pérennité de notre système de retraite et rétablir la confiance que lui portent nos concitoyens, en particulier les jeunes. Elle permettra de redonner confiance à nos concitoyens dans son équité. Aujourd'hui, compte tenu de la diversité des régimes et des règles, un euro cotisé n'ouvre pas les mêmes droits selon le statut, la forme d'emploi ou encore le profil de la carrière de l'assuré. Cette réforme permettra donc de garantir une équité de traitement entre l'ensemble des assurés. Enfin, elle devra permettre à chacun de mener des carrières nécessairement plus diversifiées qu'elles ne l'ont été dans le passé, entre statuts et régimes, sans craindre l'impact de ces choix sur ses droits à retraite. Ce projet ambitieux, nous le mènerons avec Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites, dans le cadre d'une démarche exemplaire de concertation avec l'ensemble des parties prenantes. L'ambition de transformation concerne enfin le champ de la santé. Je construis, vous le savez, la stratégie nationale de santé pour les cinq prochaines années. Je ferai connaître, en décembre prochain, les orientations précises que je retiendrai au terme de plusieurs mois de consultations et d'une grande concertation publique qui s'est ouverte mardi dernier. Ces orientations serviront de cadre à l'élaboration d'un plan national de santé et de plans régionaux de santé, au printemps. Cette stratégie privilégie quatre axes : la prévention, l'égal accès aux soins, l'innovation et la pertinence et la qualité des soins. Je souhaite évoquer d'abord la prévention, parce qu'elle est au centre de mon action. Notre système de santé est un système de soins performant. En revanche, c'est un système de prévention défaillant, à tout le moins perfectible. Les résultats médiocres que nous affichons pour certains indicateurs- je pense notamment à la mortalité avant l'âge de 65 ans -illustrent cette défaillance. C'est aussi la principale source des inégalités sociales que notre système de santé ne parvient pas à corriger. Nous devons avoir comme première priorité de changer cet état de fait, de systématiser les démarches de prévention dès le plus jeune âge, de faire en sorte qu'elles soient davantage prises en compte par les professionnels de santé dans leur pratique et que la prévention et la promotion de la santé deviennent une une part intégrante des objectifs de nos politiques publiques et des acteurs de notre société civile. Je me réjouis profondément de l'intérêt que suscite cette approche au sein de votre assemblée. Je crois que nous pouvons partager collectivement, et de façon transpartisane, dans cet hémicycle, la volonté d'un changement de méthode, d'une ambition renouvelée pour la politique de santé et même d'un réel changement de paradigme dans la conduite des politiques publiques. Ce PLFSS comporte, vous le savez, deux mesures très fortes et emblématiques de cette démarche. Nous souhaitons rendre obligatoires pour les jeunes enfants onze vaccins qui étaient jusqu'à présent, pour huit d'entre eux, simplement recommandés. Nous ne pouvons pas accepter une situation où des personnes, des enfants, sont victimes de maladies qui peuvent être évitées par la vaccination. 70 % et 80 % des enfants français reçoivent déjà ces onze vaccins. Il ne s'agit donc pas d'un bouleversement majeur des habitudes ni des attitudes vaccinales. Mais ce taux est malheureusement insuffisant pour obtenir une couverture vaccinale efficace, car il laisse la possibilité que se développent des situations épidémiques ayant des conséquences graves. Il revient donc à la puissance publique de prendre ses responsabilités. Vacciner son enfant, c'est le protéger, mais c'est aussi protéger les autres. Je veux insister sur la dimension profondément solidaire et altruiste du geste de la vaccination.

Nous avons un problème particulier avec le tabagisme : nos jeunes fument plus que dans les pays voisins et le tabagisme des femmes est particulièrement élevé en France. Le résultat, c'est près de 80 000 morts par an. Ce sont surtout des vies abrégées, des souffrances importantes que l'on pourrait éviter. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas plus de fatalité dans ces morts qu'il n'y avait de fatalité dans la mortalité sur nos routes. Le prix du tabac, c'est un fait constaté, documenté, est un paramètre important du comportement des fumeurs : il faut donc agir sur ce levier. Ce n'est bien sûr pas le seul et je ferai connaître, dans le cadre du plan national de santé, les mesures de prévention et d'incitation que je souhaite mettre en place pour aider les fumeurs à s'arrêter. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler le dialogue très constructif que j'ai eu avec Gérald Darmanin pour progresser vers cet objectif de santé publique majeur. Je veux affirmer devant vous mon égale détermination à soutenir la lutte contre les marchés parallèles, légaux ou illégaux, dans le cadre national comme dans le cadre européen, et à veiller, toujours à l'échelon européen, à la mise en place d'un système de traçabilité efficace et indépendant. L'Assemblée nationale a également souhaité, avec un soutien très large des différentes familles politiques, faire évoluer la taxation des boissons sucrées pour inciter les producteurs à réduire leur teneur en sucre. Le Gouvernement soutient cette initiative et partage le constat de l'importance d'une politique résolue et constante visant à réduire l'obésité et le surpoids. La consommation de boissons sucrées est un vecteur notable de la consommation excessive de sucre, notamment chez les plus jeunes. Il m'apparaît dès lors nécessaire et légitime de renforcer la prise de conscience collective autour des enjeux d'une alimentation équilibrée et d'inciter les acteurs de ce secteur à agir en ce sens.

Le deuxième axe de la stratégie nationale de santé concerne l'égalité d'accès aux soins. Les Français y sont légitimement très attachés, car c'est le fondement de notre modèle social. Je veux améliorer concrètement l'accès aux soins. Les difficultés sont d'abord liées au montant des restes à charge. C'est en particulier vrai, de longue date, dans trois domaines du soin : l'optique, le dentaire et les audioprothèses, où l'assurance maladie couvre moins bien la dépense, où les assureurs complémentaires ont parfois pris le relais, mais où, globalement, le reste à charge pour le patient est très élevé. Cette situation est le fruit de l'histoire, d'arbitrages successifs qui ont conduit à créer des « angles morts » de la protection sociale, pour des soins ou des prestations qui rendent pourtant un service important aux patients et réduisent le risque de « bascule » dans la dépendance. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'il en soit toujours ainsi. C'est pourquoi j'ai commencé le travail et la concertation pour aboutir à un reste à charge « zéro » dans les domaines de l'optique et des audioprothèses, en sus des négociations entamées à la mi-septembre dans le secteur dentaire. Ces travaux devront aboutir, en tout état de cause, avant la fin du premier semestre de 2018. Permettez-moi, dans ce contexte, d'évoquer le tiers payant. Vous le savez, le récent rapport que l'IGAS- l'Inspection a conclu que la généralisation du tiers payant à la date du 30 novembre prochain, telle que la prévoyait la loi du 26 janvier 2016, était irréaliste. J'en ai tiré les conclusions en proposant au Parlement de lever cette obligation. Le tiers payant restera bien entendu obligatoire là où il s'applique déjà et où il fonctionne bien, c'est-à-dire pour les personnes souffrant d'une affection de longue durée, ou ALD, prise en charge à 100 %, pour les femmes enceintes ou pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, la Mais je veux vous dire également mon attachement à ce que le tiers payant se généralise pour les consultations médicales, comme cela a été le cas pour les médicaments, et ma détermination à faire aboutir les travaux qui permettront de rendre le système simple d'utilisation pour les professionnels. Le Gouvernement s'est engagé à présenter au Parlement, d'ici au 31 mars 2018, un calendrier de déploiement opérationnel du tiers payant intégral dans des conditions techniques fiabilisées. À cette date, nous identifierons également des publics prioritaires, au-delà des publics déjà couverts, pour lesquels un accès effectif au tiers payant intégral devrait être garanti. Nos concitoyens sont également de plus en plus préoccupés par l'égal accès aux soins sur le territoire, et je sais la Haute Assemblée fortement mobilisée sur cette question. J'ai présenté, le 13 septembre dernier, avec le Premier ministre, un plan pour renforcer l'égal accès aux soins. Le constat que nous pouvons faire, c'est que nous n'avons pas su assez anticiper l'évolution de l'exercice médical, des attentes des nouvelles générations de médecins et surtout le fait que l'évolution du profil des patients nécessite une prise en charge par des équipes de soins composées du médecin et d'autres professionnels de santé. Je ne crois ni la coercition ni à l'obligation. Il n'y a pas une solution unique aux difficultés que rencontrent nos concitoyens, mais des solutions, adaptées à chaque territoire, et portées par les acteurs de terrain.

libérer du temps médical en levant les freins administratifs, notamment en favorisant le cumul emploi-retraite, les remplacements, les consultations avancées et l'exercice coordonné sous toutes ses formes. est le sens du plan d'action que nous avons bâti et qui devra continuer à être enrichi, avec la contribution des élus, au cours de la mandature. En appui de ce plan, le projet la généralisation de l'usage de la téléconsultation et de la téléexpertise, en les sortant de leur cadre expérimental. S'agissant maintenant de l'innovation et de la pertinence des soins, je veux en particulier faciliter l'expérimentation de formes nouvelles d'organisation et de rémunération. Elles Elles permettront de dépasser les logiques sectorielles ville-hôpital, de rémunérer par exemple au forfait des séquences de soins, de prendre en compte la prévention, ainsi que la pertinence des actes réalisés. Je vous proposerai donc d'adopter, à l'article 35 de ce projet de loi, un cadre général, valable pour le quinquennat, qui permettra de lancer et d'évaluer ces expérimentations. ces expérimentations. Elles pourront être financées par un fonds d'innovation qui sera abondé en tant que de besoin par l'assurance maladie. Mon objectif, à terme, est bien de faire évoluer et de compléter les dispositifs actuels de rémunération, à savoir la rémunération à l'acte et la tarification à l'activité. Je suis en effet convaincue que le levier tarifaire est un levier fondamental de l'évolution de notre système de santé vers plus de prévention, de coopération entre professionnels et de pertinence des soins.

Je veux vous dire ma disponibilité pour travailler de concert à ce que les professionnels et les organisations prennent mieux en compte cet objectif. Je veux terminer en évoquant l'évolution de la dépense d'assurance maladie, et Il sera fixé à 2,3 %. Ce taux est conforme à l'engagement du Président de la République. Il est supérieur à celui des trois années précédentes et permettra de consacrer 4,4 milliards d'euros supplémentaires à la couverture des soins.

C'est pourquoi le sous-objectif des soins de ville, fixé à 2,4 %, sera supérieur au taux global de l'ONDAM. J'estime que cette convention va dans le sens des orientations que je porte : elle valorise mieux l'action des généralistes et prend mieux en compte, notamment, les actes complexes ou réalisés dans des situations d'urgence. L'évolution des ressources des établissements de santé sera fixée pour sa part à 2,2 %, du fait de l'apport que constituera pour les établissements de santé le relèvement de 2 euros du forfait journalier. 400 millions d'euros seront dédiés à l'investissement immobilier et numérique. Près de 600 millions d'euros seront consacrés à l'augmentation des dépenses de la liste en sus, liée à l'arrivée des nouvelles classes thérapeutiques innovantes. plus de 200 millions d'euros, permettront de mettre en oeuvre des actions indispensables dans le cadre de nos politiques publiques, visant notamment à mieux faciliter l'accès aux soins des populations précaires. Enfin, le Fonds d'intervention régional, le FIR, sera augmenté de 3,1 %. Il doit être, avec le fonds d'innovation que j'évoquais précédemment, le support d'une politique de transformation au plus près du terrain. Un taux d'ONDAM de 2,3 % reste un taux exigeant. Cela doit nous inviter à poursuivre la réorganisation de notre offre de soins et à orienter toujours plus notre offre de santé vers la pertinence : plusieurs dispositions du projet de loi de financement Nous devons également, pour les prestations de santé comme sur l'ensemble du champ de la sécurité sociale, être vigilants pour détecter et juguler la fraude. Nous avons formulé des propositions en ce

Donner des perspectives, c'est engager des réformes en profondeur et bouger les lignes pour faire progresser notre collectivité nationale. La parole

qu'il s'agisse des ressources de la protection sociale, de son organisation ou des défis à relever pour la moderniser dans la période qui s'ouvre, ce premier projet de loi de financement de la sécurité sociale du quinquennat est porteur de réformes significatives. Nous attendons avec intérêt, madame la ministre, les projets que vous avez évoqués concernant l'accès aux soins et, notamment, la réforme des retraites. Face à l'allongement de l'espérance de vie, au vieillissement, à la dépendance, au développement des maladies chroniques, mais aussi des thérapies personnalisées et des prises en charge innovantes, nous ne pourrons plus injecter de nouvelles recettes sans mettre à mal le pouvoir d'achat des actifs et la compétitivité des entreprises. C'est donc dans la pertinence des actes et des prises en charge, dans la maîtrise médicalisée des dépenses, dans la recherche du meilleur soin au meilleur coût et au bon moment pour le patient que nous trouverons les ressources nécessaires pour faire de la place à l'innovation et aux besoins sociaux de la population. Le dossier médical partagé, le DMP, tant attendu, pourra y contribuer. Le Sénat tient ce discours, et le répète, depuis longtemps. Je suis heureux, madame la ministre, de le voir enfin entendu, lorsque vous reprenez à votre compte l'impératif de la lutte contre les actes inutiles. Enfin, la politique du rabot, qui nuit tant à nos hôpitaux, cède la place à la recherche de l'efficience ! Bien sûr, c'est plus difficile, cela bouscule un peu les positions acquises. vous nous trouverez à vos côtés dans cet engagement, parce que c'est l'avenir de notre système de protection sociale, au coeur de l'identité de notre pays, qui est en jeu. La stratégie de santé que vous proposez affiche une autre priorité, la prévention. Nous trouvons, notamment sociale, des taxes comportementales sur le tabac et les boissons sucrées, qui répondent à cet objectif et que nous approuvons. Pour ce qui concerne les ressources de la sécurité sociale, la CSG est réaffirmée comme l'impôt de la protection sociale, en substitut de cotisations salariales, avec, à la clé, pour les actifs, plusieurs milliards d'euros de gains de pouvoir d'achat. Notre commission partage le constat selon lequel il convient de diversifier les recettes de la sécurité sociale, afin que son coût ne repose pas uniquement sur le travail. Mais cette réforme a été mal expliquée et, par conséquent, mal comprise. Seule l'augmentation de la CSG a été retenue parmi les annonces, en raison, notamment, du sort fait à certaines catégories de retraités, qui ne bénéficient ni de l'exonération ni du taux réduit. À titre personnel, je l'ai dit en commission des affaires sociales, je ne suis pas hostile à une convergence progressive de la CSG des retraités et des actifs, dans la mesure où les niveaux de vie sont aujourd'hui comparables. Mais cette hausse n'est pas une convergence ; elle est perçue comme injuste et punitive, notamment pour les tranches supérieures, lesquelles ne bénéficieront d'aucune C'est pourquoi la commission des affaires sociales a marqué son opposition à cette mesure, et vous engage à explorer d'autres pistes, moins stigmatisantes. Après les ménages, le texte s'adresse aussi aux entreprises, avec la baisse des cotisations pour les indépendants, l'année blanche pour les créations d'entreprises et la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, en réduction de cotisations sociales. Cette dernière s'opère par une réduction de 6 points du taux de cotisation maladie jusqu'à 2,5 SMIC. Le coût de cette mesure serait de 21,6 milliards d'euros. Elle se traduit également par un approfondissement des allégements généraux de cotisations au voisinage du SMIC, qui concernerait les contributions patronales d'assurance chômage et les cotisations aux régimes complémentaires Au niveau du SMIC, les cotisations seraient donc résiduelles. Cet approfondissement des allégements généraux représente 3,3 milliards En 2019, les entreprises bénéficieront donc du versement du CICE dû au titre de 2018 et des réductions de cotisations, ce qui représente un effort plus que significatif. Pour les entités bénéficiaires du crédit d'impôt de taxe sur les salaires, le CITS,- je pense notamment à l'aide à domicile -, le gain est de 800 millions d'euros. Le positionnement des allégements sur les bas salaires a paradoxalement donné lieu à peu de débats, alors que les effets sectoriels de ces choix ne sont pas négligeables : les allégements généraux sur les bas salaires bénéficient prioritairement à des entreprises de petite taille, dans des secteurs peu exposés à la concurrence internationale. Ils ne profitent que faiblement à l'industrie. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est exprimé sur la nécessité de réfléchir aux prélèvements sociaux sur les salaires plus élevés, et notre commission souhaite que ce débat soit ouvert. La transformation du CICE nous offre l'occasion de revisiter toute une série de dispositifs sectoriels de réductions de cotisations. La réduction des fameuses « niches sociales » est un serpent de mer, et les tentatives, anciennes ou récentes, se sont soldées par des échecs le cadre général étant désormais très incitatif sur les bas salaires, il serait souhaitable qu'elle aboutisse enfin. S'agissant de la protection sociale des travailleurs indépendants, la commission des affaires sociales a pris acte du principe de l'intégration du RSI au régime général,

Il faut apprendre de celles du passé ! Cette réforme exige un portage politique sans relâche, des systèmes d'information efficaces et, surtout, une attention constante aux acteurs de cette protection sociale, qu'il s'agisse des salariés du régime ou des indépendants, aux attentes légitimes. Pour reprendre les mots de nos collègues Jean-Noël Cardoux et Jean-Pierre Godefroy, il faut restaurer la confiance. Vous trouverez notre commission vigilante sur ce dossier. Elle a adopté plusieurs amendements, qui soulèvent autant de questions sur lesquelles nous souhaitons que vous puissiez vous engager l'accueil des travailleurs indépendants dans le nouveau schéma, le pilotage de la réforme, les systèmes d'information ou encore l'assiette des cotisations et leur paiement. S'il est une population pour laquelle le prélèvement à la source a du sens, ce sont bien les travailleurs indépendants, dont les revenus se caractérisent par une forte volatilité. Il faut traiter ces questions, faute de quoi la réforme passera à côté des sujets de préoccupation des indépendants et risque de décevoir. Plus encore, elle est le test de la capacité de ce gouvernement à réformer notre protection sociale. Nous n'oublions pas que se profile ensuite la réforme des retraites. Ces différentes réformes et la perspective d'un retour à l'équilibre des comptes sociaux ne doivent pas faire oublier les déficits passés, qui représenteront 21,3 milliards d'euros, portés par l'ACOSS, l'Agence

Les montants en jeu sont importants, alors que l'équilibre n'est pas acquis. Ils sont portés en trésorerie et potentiellement exposés à l'augmentation des taux d'intérêt à court terme. concerne cette dette, les intentions du Gouvernement sont à clarifier. Il a été indiqué devant notre commission que les excédents futurs des différentes branches viendraient la résorber à partir de 2019. Dans le même temps, le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit le plafonnement de l'excédent des comptes sociaux à partir de 2019, légèrement au-dessus du niveau de l'amortissement opéré par la CADES, dont le montant s'élève encore à 131 milliards d'euros. Ainsi pour résorber la dette supplémentaire de l'ACOSS. Notre commission s'interroge très fortement sur l'opportunité d'une telle démarche, et même sur sa rationalité économique. La dette sociale est une anomalie qu'il convient de faire disparaître au plus vite. Si notre commission est tout à fait prête à un débat sur les relations financières entre l'État et la sécurité sociale, le maintien de la dette sociale à court terme, en raison du transfert à l'État des excédents sociaux, ne lui paraît pas de bonne politique. Telles sont les principales observations que je souhaitais faire, au nom de la commission des affaires sociales, sur ce PLFSS. Dans la crise de défiance que nous vivons, il faut faire la démonstration de notre capacité à retrouver et à conserver l'équilibre des comptes sociaux, à assurer la pérennité du système de retraite, grâce à la réforme systémique que le Sénat appelle de ses voeux, et à garantir la transparence et l'équité du système de soins. sociale trace quelques pistes, forcément insuffisantes, parfois risquées, encore à consolider, mais que notre commission souhaite encourager.

Elle porte également une part prépondérante du déficit des comptes sociaux. Dans ce contexte, la trajectoire de retour à l'équilibre de la branche est un objectif que, bien entendu, nous partageons, bien qu'il s'agisse, nous le savons, d'un objectif exigeant. Il implique, dans la durée, des changements plus profonds que de simples ajustements, vécus chaque année dans la tension par les acteurs du système de santé. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale laisse, à cet égard, nombre d'observateurs interrogatifs, tant les attentes sont fortes. Sans que le texte traduise encore des choix stratégiques, la commission des affaires sociales a estimé qu'il présentait, s'agissant de la branche maladie, des inflexions positives. Elle a ainsi salué l'accent porté sur la prévention, l'innovation et la pertinence des soins. Elle a apporté son soutien à l'extension de la vaccination obligatoire des jeunes enfants, comme au renforcement de la fiscalité du tabac. Elle a également approuvé le cadre expérimental pour l'innovation et le déploiement tant attendu de la télémédecine, qui apportera une réponse - ce ne sera pas la seule - aux enjeux de l'accès aux soins. Notre système de santé ne se transformera pas sans la confiance de ses acteurs de terrain et, en premier lieu, des professionnels de santé. Les expérimentations devront offrir un cadre souple, associer l'ensemble des acteurs, soutenir les initiatives locales, pour déboucher, nous le souhaitons, sur des évolutions pérennes. Tel est le sens de plusieurs amendements que je présenterai. Dans le même objectif d'accompagnement de l'innovation, la commission a souhaité rétablir la procédure accélérée d'inscription des actes à la nomenclature, tout en préservant le rôle dévolu aux professionnels de santé. Elle a aussi regretté que les enjeux de l'accès précoce des malades aux traitements innovants soient absents du texte. Des adaptations du dispositif des autorisations temporaires d'utilisation, les ATU, sont souhaitées par les professionnels médicaux, en particulier pour faciliter les extensions d'indications. Les règles de recevabilité financière ne me permettent pas de proposer une telle évolution. Toutefois, je présenterai un ajustement plus technique sur cette question. Madame la ministre, pourrez-vous nous préciser vos intentions sur ce sujet, qui mériterait, me semble-t-il, une remise à plat globale ? En ce qui concerne la maîtrise des dépenses de santé, la commission apprécie et soutient l'approche fondée sur la pertinence des soins. Cependant, sa traduction dans le texte demeure encore trop partielle et, parfois, discutable. S'agissant ainsi de la régulation du dispositif médical, la commission a jugé nécessaire d'adapter les mesures proposées à la réalité de ce secteur économique, car il est important de ne pas fragiliser le tissu des petites entreprises.

La commission salue, madame la ministre, votre décision pragmatique sur le tiers payant. Sachez que nous restons opposés à toute obligation au-delà des publics prioritaires. La confiance des professionnels de santé est aussi en jeu dans les discussions en cours avec les chirurgiens-dentistes. Vous savez notre attachement à la négociation conventionnelle. La commission a validé le report du règlement arbitral, à laquelle elle s'était toujours opposée, mais elle sera attentive à ce que les engagements pris soient tenus. Pourrez-vous nous donner, madame la ministre, au cours des débats, des assurances à ce sujet ? Enfin, le plan que vous avez annoncé en faveur de l'accès aux soins est très attendu dans nos territoires. Je souhaite à cet égard attirer votre attention sur les complémentarités nécessaires entre les établissements publics et privés de santé. La possibilité, pour ces derniers, de se voir confier des missions de service public serait une reconnaissance fortement attendue de leur rôle dans l'offre de soins. Pourrez-vous nous faire part de vos orientations sur cette question ?

c'est avec honneur et gravité que je rapporte pour la première fois devant vous les crédits consacrés par l'assurance maladie au financement du secteur médico-social. Les chiffres peuvent paraître satisfaisants. Un ONDAM médico-social à 20,5 milliards d'euros, en progression de 2 % par rapport à 2017, confirme l'effort entrepris en faveur des publics handicapés et en perte d'autonomie. Les autres produits affectés au financement des dépenses de soins en établissement, essentiellement de nature fiscale, ne peuvent faire l'objet de la même prévision, mais on anticipe pour l'ensemble de ces dépenses un montant global de 22 milliards d'euros en 2018. Le Sénat maintiendra sa vigilance quant au suivi de ces dotations. Trop de mesures nouvelles ont été annoncées sans connaître de réalisation effective au cours des exercices précédents pour que nous placions une confiance aveugle dans les 515 millions d'euros supplémentaires promis par le Gouvernement. Nous serons attentifs à ce que les plans de création de places voient le jour et que leur lancement subisse moins d'entraves administratives. Certes, le Gouvernement y veille en partie par l'introduction de la caducité partielle, mais nous devrons pousser plus loin la réflexion en questionnant en profondeur le modèle des appels à projets et l'extension de leur champ d'exonération. La restructuration de l'offre médico-sociale est l'un des plus grands défis de ces prochaines années. C'est un chantier engagé depuis quelques années par des gouvernements qui ont rénové par retouches successives les modes de tarification des établissements, soumettant certains d'entre eux, ainsi que leur régime contractuel, Ces réformes, qui approfondissent la responsabilisation des gestionnaires, vont dans le bon sens ; nous les accueillons favorablement. Mais nous aurions préféré qu'elles fassent l'objet d'une concertation préalable de grande ampleur, les acteurs des secteurs du grand âge et du handicap, plutôt que d'être glissées par fragments, de PLFSS en PLFSS, sans qu'aucun discours pédagogique vienne rassurer les gestionnaires ou les familles. L'attention très récemment portée par les médias à ces questions ne vous a-t-elle pas convaincue, madame la ministre, de l'impérieuse nécessité de parler, de partager, de communiquer sur ces réformes, au lieu de les concevoir dans l'ombre des cabinets et des administrations ? âgées dépendantes, qui sont dans l'inquiétude. Nombre d'entre eux, particulièrement au sein du secteur public, s'estiment lésés par la réforme de la dotation à l'autonomie, conduite dans une opacité regrettable s'agissant de mesures en apparence paramétriques, mais aux incidences bien réelles. Ce n'est que cet été que les acteurs de la prise en charge du grand âge ont pris conscience des retombées fâcheuses qu'un décret de décembre 2016 pouvait avoir sur leur budget. Entre-temps, les enquêtes menées par vos services ont apporté quelques éléments susceptibles de les rassurer ; quelques défauts méthodologiques ont néanmoins été soulevés et la représentation nationale ne s'estime pas totalement apaisée sur ce point. Pouvez-vous réaffirmer aujourd'hui devant nous, madame la ministre, que les pertes subies par les EHPAD publics seront intégralement couvertes par les financements d'appui de 28 millions d'euros que vous annoncez ? Pouvez-vous garantir que cette réforme ne nous fera pas à terme courir le risque d'une déshabilitation massive à l'aide sociale ? La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité, pour sa part, contribuer à la lisibilité de la réforme de l'offre médico-sociale, en accompagnant le mouvement de contractualisation pluriannuelle et en sécurisant le régime de la caducité partielle.

malgré de nouvelles dépenses mises à sa charge, le solde prévisionnel de la branche s'élèverait à 500 millions d'euros en 2018. Ce résultat est d'autant plus remarquable que son financement repose intégralement, je le répète, qui ont consenti des efforts répétés ces dernières années pour apurer la dette. Car celle-ci, je le rappelle, ne fait pas l'objet de reprises par la CADES, contrairement à ce qui s'est passé Compte tenu de cette situation, nous regrettons que les mesures nouvelles pour la branche AT-MP demeurent finalement assez timides, même s'il s'agit d'avancées auxquelles nous ne pouvons qu'être favorables et même si les résultats obtenus en matière de sinistralité sont très encourageants.

Une partie grandissante des ressources de la branche AT-MP est en fait consacrée à des transferts vers d'autres branches ou vers des fonds. Elle est en particulier le principal financeur des dispositifs mis en place pour les victimes de l'amiante,

À lui seul, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, a été doté de 5,6 milliards d'euros depuis sa création, dont 5,1 milliards d'euros en provenance de la branche AT-MP. Pour la première fois, les dépenses d'indemnisation ont connu en 2016 une baisse, que l'exercice 2017 semble confirmer. Vingt ans après le début de l'interdiction de l'usage de l'amiante, une telle inflexion pourrait indiquer le passage d'un cap compte tenu du délai de latence des maladies liées à l'amiante, les études épidémiologiques prévoyaient un pic des demandes en 2020. Avec une légère avance par rapport aux prévisions, ce pic pourrait donc être aujourd'hui dépassé, ce qui est encourageant. La situation du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le FCAATA,

l'information des personnes ayant demandé l'inscription d'un établissement sur la liste des employeurs ouvrant droit à l'ACAATA, l'allocation de cessation

Au total, les dépenses de la branche AT-MP au titre des fonds Amiante ont désormais plutôt tendance à diminuer. Tel n'est pas le cas des dépenses durablement générées pour la branche par la réforme du compte pénibilité, le 1 octobre dernier.

Il semble d'ailleurs que la CNAMTS ait pris connaissance assez tardivement du transfert envisagé par le Gouvernement ; l'évaluation de l'impact financier de la mesure demeure peu approfondie. La branche sera probablement confrontée à une hausse importante des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles. En outre, si la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, avait mis en place un dispositif d'ouverture et de gestion des droits, elle n'avait pas développé l'activité de prévention en entreprise. Tout l'enjeu sera d'y affecter les moyens nécessaires et d'éviter de rester dans une simple logique de réparation. Dans ce domaine, madame la ministre, veillons à ce que les efforts d'économies demandés à la branche AT-MP de la CNAMTS n'obèrent pas sa capacité d'action. Enfin, notre commission s'interroge une nouvelle fois sur l'avenir du versement à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des AT-MP. Ce transfert, qui s'élève à 1 milliard d'euros, ce qui n'est pas rien, est entièrement financé par des ressources mutualisées entre les employeurs. Les limites de l'exercice d'évaluation, qui débouche sur un mécanisme par nature inflationniste, sont connues. En outre, au regard de la progression continue du transfert, il est permis de s'interroger sur la réalité des efforts engagés pour lutter contre la sous-déclaration. Au-delà de 2018, le PLFSS prévoit la poursuite de la croissance des excédents de la branche AT-MP. Il paraît légitime d'en tirer les conséquences pour les employeurs, en engageant une décroissance des taux de cotisation. Il nous faudra cependant être vigilants concernant l'avenir des dépenses mutualisées, afin d'éviter qu'elles ne fragilisent les fondements assurantiels de ce système centenaire, qui a su s'adapter aux évolutions de la société et auquel notre commission des affaires sociales a toujours été très attachée.

Mme la ministre, au nom de la commission des affaires sociales. La première concerne la dégradation des perspectives financières du système de retraites. À l'horizon de 2021, le solde des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse,

Après la présentation abusivement optimiste des comptes l'an dernier, ce PLFSS remet les pendules à l'heure. Il dévoile un besoin de financement qui, sans être catastrophique, n'en demeure pas moins, me semble-t-il, inacceptable pour les générations futures, futures, d'autant que les dernières projections du Conseil d'orientation des retraites, le COR, montrent qu'à réglementation inchangée, le système de retraites demeurerait déficitaire

Enfin, le comité de suivi des retraites a, pour la première fois depuis sa création, recommandé au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ramener le système de retraites sur une trajectoire d'équilibre. Aucune mesure de ce PLFSS ne répond à l'enjeu financier, excepté le nouveau décalage de la revalorisation des pensions, qui ferait économiser environ 340 millions d'euros en 2018.

le Sénat avait proposé de porter à 63 ans l'âge légal de départ, et d'accompagner ainsi l'accord courageux des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO signé en 2015. Nous prêchions à l'époque dans le désert. Qu'en sera-t-il sous ce quinquennat ? deuxième source d'inquiétude, madame la ministre, concerne le Fonds de solidarité vieillesse, dont le Sénat a suivi de près les évolutions grâce à ses rapporteurs de renom, Gérard Roche et Catherine Génisson. Les gouvernements successifs se sont accommodés du déficit de ce fonds, modifiant d'année en année ses recettes ou ses charges, à la faveur d'un jeu de tuyauterie habituel en matière de sécurité sociale. En 2018, il affichera encore un déficit de 3,4 milliards d'euros, proche de ceux de 2016 et de 2017, alors même que la dernière loi de financement de la sécurité sociale, en lui retirant progressivement le financement du minimum contributif, le MICO, allégeait ses charges de 1 milliard 2017 et de près de 800 millions d'euros supplémentaires pour 2018. Deux dispositions nous laissent craindre que votre gouvernement, madame la ministre, n'utilise lui aussi le FSV comme un agent de trésorerie des régimes de retraite.

Ainsi, l'une des mesures phares du Président de la République à destination des retraités les plus modestes n'est tout simplement pas financée, ou l'est par la dette ! Quant à la dette du FSV, portée par l'ACOSS, elle se creuse : 11 milliards d'euros en 2018, plus de 15 milliards en 2021.

l'effort actuellement demandé aux retraités est substantiel. Mettre les retraités à contribution constitue l'un des trois leviers classiques pour équilibrer les retraites, avec la hausse des cotisations et l'allongement de l'activité. L'orientation prise dans ce PLFSS augure-t-elle des choix à venir au titre de la réforme des retraites ?

Attachée, comme nombre d'entre vous, à notre modèle de politique familiale, je ne peux,, que me réjouir de cette situation. Pour autant, les conditions de ce retour à l'équilibre suscitent Si le redressement des comptes de la branche résulte, en partie, de l'amélioration de la conjoncture économique et d'un transfert de charges vers l'État, il est aussi le fruit d'importantes mesures d'économies. L'impact de l'ensemble des réformes intervenues dans le champ de la politique familiale depuis 2012 s'élève environ, cette année, à 1,5 milliard d'euros d'économies, assumées par les familles. La majeure partie de ces efforts a été supportée par des familles relativement aisées, au travers des abaissements du plafond du quotient familial et de la modulation des allocations familiales. Pour autant, les familles des classes moyennes n'ont pas été épargnées par les mesures portant sur des prestations sous conditions de ressources. Au-delà de ce rabotage, qui est préoccupant dans un contexte de baisse du nombre des naissances, l'évolution de la politique familiale au cours de la période récente nous interpelle. Elle remet en effet en cause quelques-uns des principes fondateurs de cette politique, alors même que certains de nos voisins souhaiteraient aujourd'hui s'en inspirer. inspirer. La politique familiale a été conçue dans une logique de compensation des charges de famille et de solidarité horizontale. Si des aides spécifiques ont été instaurées en faveur de publics ciblés, la notion d'universalité demeurait centrale. En supprimant presque intégralement les prestations d'entretien dont bénéficient les familles aisées et en resserrant les montants et les conditions de ressources des prestations destinées aux classes moyennes, les mesures prises durant le quinquennat précédent ont réorienté la politique familiale vers la lutte contre la pauvreté. Cette évolution, qui a parfois semblé résulter davantage d'une succession de mesures d'économie que d'une orientation assumée, pose un certain nombre de questions. Doit-on renoncer au principe de compensation des charges de famille et aider uniquement les familles exposées au risque de pauvreté ? À revenus équivalents, une famille aisée avec enfants a-t-elle droit à davantage d'aides qu'un couple sans enfant ? Quelle serait l'acceptabilité sociale d'une politique familiale excluant de ses bénéfices ses principaux financeurs ? doit-elle être étendue à d'autres domaines, comme l'assurance maladie, voire l'accès aux services publics ? Alors que s'ouvre un nouveau quinquennat et qu'une nouvelle convention d'objectifs et de gestion doit être conclue entre l'État et la CNAF, il convient donc de définir la place que nous souhaitons collectivement accorder aux familles dans notre modèle de société. Madame la ministre, j'ai bien entendu votre volonté de donner du sens à la politique familiale.

L'augmentation des plafonds de prise en charge au titre du complément de libre choix du mode de garde pour les familles monoparentales est relativement consensuelle. Il s'agit d'aider davantage un public, majoritairement féminin, qui est particulièrement touché par la pauvreté et l'éloignement du marché du travail. Pour autant, il ne faut pas exagérer sa portée. Le coût de cette mesure, 40 millions d'euros en année pleine, indique que le bénéfice pour les familles concernées sera nettement moins important que les montants théoriques présentés par l'étude d'impact. À l'inverse, l'alignement par le bas des montants et plafonds de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE, sur ceux du complément familial représente une économie qui atteindrait à terme 500 millions d'euros par an.

Les justifications avancées par le Gouvernement ne font pas disparaître le sentiment que les prestations familiales sont utilisées comme variables d'ajustement budgétaire, dans la continuité de la période précédente. Nous reviendrons sur ce point au cours des débats sur l'article 26, que la commission des affaires sociales vous proposera de supprimer, mes chers collègues. Sous cette réserve, et tout en soulignant que ce PLFSS ne traite pas les défis auxquels la politique familiale fait face, la commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'objectif des dépenses de la branche famille. Mais le débat est ouvert, et nous y participerons avec plaisir

notamment des transferts financiers entre le budget de la sécurité sociale et celui de l'État ou du « poids » des administrations de sécurité sociale dans les finances publiques. À ce titre, le Gouvernement compte principalement sur les administrations de sécurité sociale pour atteindre l'objectif de ramener le déficit public

près de la moitié des économies à réaliser d'ici à 2022 reposent sur les administrations de sécurité sociale. C'est beaucoup, madame la ministre ! Il s'agit d'un pari risqué. Compte tenu des mesures proposées pour 2018, qui reposent sur des leviers traditionnels déjà largement exploités, il est permis de douter de l'objectif que le Gouvernement s'est fixé d'un retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale à l'horizon de 2020. Je souhaiterais d'abord revenir sur la modification structurelle du financement de la sécurité sociale proposée par le Gouvernement et sur la suppression du CICE, qui sera transformé en baisse de charges

laquelle s'ajoutera au gel des pensions de retraite en 2018, « année blanche » résultant du report de la revalorisation des pensions. La commission des finances a donc adopté un amendement supprimer la hausse de la CSG pour les 60 % de personnes retraitées qui auraient été concernées par cette augmentation. La transformation proposée du CICE en baisse de cotisations patronales est une autre avancée positive.

maintenant aux choix du Gouvernement en matière de maîtrise de la dépense sociale, qui conduisent à douter de la trajectoire annoncée des comptes sociaux. En recettes, la réduction prévue des déficits repose sur le dynamisme des recettes,

sur ces deux branches, des dépenses nouvelles sont annoncées par le Gouvernement, mais sont en réalité plus que compensées par de nouvelles mesures d'économies. Le revalorisation du minimum vieillesse coûtera 115 millions d'euros en 2018 ; « en même temps », l'alignement des revalorisations des pensions de retraite et du minimum vieillesse au 1 janvier conduit à un gel des pensions de retraite qui permet d'économiser 380 millions d'euros en 2018,

Un couple d'instituteurs, par exemple, perdrait près de 2 000 euros d'allocations l'année suivant la naissance de son premier enfant ! Voilà une nouvelle économie, de 500 millions d'euros par an à compter de 2022, réalisée cette fois sur le dos des familles.

de motifs d'inquiétude sur les conditions de rattachement des indépendants au régime général, mais aussi de vraies satisfactions, en particulier sur le volet « santé ». Après un quinquennat dont nous ne partagions pas les choix, cette appréciation nuancée traduit néanmoins une certaine déception. Globalement, à la faveur de meilleures perspectives économiques, le déficit de la sécurité sociale s'atténue, sans qu'il soit besoin de recourir, comme l'an passé, à de multiples artifices de présentation. Ce déficit pourrait même faire place, d'ici deux ans si les hypothèses se vérifient, à des excédents. C'est visiblement sur ces excédents que compte le Gouvernement pour apurer la dette d'une vingtaine de milliards d'euros qui reste aujourd'hui gérée en trésorerie par l'ACOSS. La branche famille est excédentaire, mais c'est au prix de mesures que le Sénat avait dénoncées, et l'économie sur la PAJE, prévue à partir de l'an prochain, nous semble injustifiée. Madame la ministre, devant notre commission, vous avez indiqué vouloir mener un débat « apaisé » sur l'avenir de notre politique familiale. Mais s'il en résultait de nouveau la réduction de toute forme de compensation des charges familiales au-delà d'un certain niveau de revenu, cela viderait de sa substance une politique dont la réussite tenait au profond sentiment qu'elle s'adressait à tous, sans exception. de la branche vieillesse, le déficit repart à la hausse. Je n'insiste pas, car nous avions absolument contesté, l'an dernier, l'idée selon laquelle le problème des retraites aurait été réglé. Il s'agit donc d'un retour à la réalité, sans pour autant que le Gouvernement, pour l'instant, en tire de conséquence.

Il faudra donc y répondre rapidement, sans attendre une future modification de l'architecture et des paramètres des différents régimes, d'autant que l'exercice sera nécessairement complexe à mener.

et non d'un simple article soumis au Parlement dans les délais d'examen très brefs propres au PLFSS. Sur l'assurance maladie, la commission des affaires sociales porte une appréciation plus positive. Nous soutenons pleinement les mesures sur le tabac, la vaccination, les consultations de prévention pour les jeunes femmes. La suppression de l'obligation générale du tiers payant témoigne d'un changement d'approche indispensable vis-à-vis des professionnels de santé. Enfin, nous approuvons les mesures en faveur de nouvelles formes de prise en charge. Sans doute ne seront-elles pas suffisantes pour donner corps à cette ambition que nous partageons avec vous,

comme on le constate notamment dans les établissements hospitaliers. Si j'ai parlé il y a quelques instants de déception, c'est que, sur la question essentielle du financement, je ne vois pas clairement où nous mènent les choix opérés par le Gouvernement ; je ressens même, en la matière, La principale mesure du programme de législature réside dans la hausse de la CSG au 1 janvier prochain. De cette mesure, il ne résulte ni ressources supplémentaires pour la sécurité sociale ni baisse du coût du travail. Assortie de multiples compensations, dont toutes, à ce jour, ne sont pas arrêtées, elle entraîne un gain de pouvoir d'achat pour une majorité d'actifs et une perte pour beaucoup de retraités. Elle s'accompagne de complexes circuits de transferts, entre l'État et la sécurité sociale comme au sein de celle-ci. Tout cela, de mon point de vue, brouille plus qu'il ne clarifie le financement de la protection sociale. C'est aussi la première fois, me semble-t-il, qu'on touche aux cotisations d'assurance chômage au sein d'un PLFSS. Cette première sera peut-être aussi une dernière, puisque l'exonération prévue équivaut à une suppression pure et simple de la part salariale. Le plus étonnant est que cette modification du financement de l'assurance chômage s'opère alors que les discussions sur sa future réforme ne sont pas encore engagées. Nous ignorons aujourd'hui ce qu'il en sera de l'extension aux démissionnaires et aux indépendants, ainsi que du financement d'une telle réforme et de ses implications sur la gestion paritaire de l'UNEDIC. Madame la ministre, pourquoi ne pas avoir attendu un an de plus pour nous présenter un projet cohérent sur la couverture des différents risques et les ressources qui en garantiront le financement ? La hausse de la CSG renforce la part de l'impôt dans le financement de la sécurité sociale, alors que cette dernière ne recevra pratiquement plus de TVA de la part de l'État. En définitive, la sécurité sociale sollicitera davantage les revenus d'activité et moins la consommation.

Cette mesure nous éloigne également un peu plus du principe selon lequel les impôts financent la solidarité et les cotisations les risques assurantiels. Enfin, il me paraît nécessaire de préserver la spécificité des finances sociales. C'est d'ailleurs l'un des grands acquis de la réforme constitutionnelle de 1996. Ses auteurs ont voulu que le Parlement se prononce sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale, de manière à discuter dans un ensemble cohérent du niveau de couverture sociale de nos concitoyens et des ressources que la collectivité y consacre. La semaine dernière, nous examinions un projet de loi de programmation quinquennale qui annonçait une remise en cause à venir de la compensation par l'État des exonérations de cotisations sociales. Avec la hausse de la CSG et les mesures qui l'accompagnent s'amorce déjà un déséquilibre des relations financières entre l'État et la sécurité sociale. En supprimant la hausse de la CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité, la commission des affaires sociales a voulu corriger le point le moins acceptable à ses yeux du volet « recettes » du PLFSS. Mais, au-delà de cet aspect particulier, je reste réservé sur l'orientation qui semble se dessiner en matière de financement de la protection sociale, ce qui ne m'empêche pas de reconnaître par ailleurs, dans le domaine de la politique de santé notamment, plusieurs mesures positives de ce PLFSS. Nous passons

c'est un autre projet de loi de financement de la sécurité sociale que nous vous invitons à écrire, dégagé de la mainmise étatique que le Gouvernement veut imposer à la sécurité sociale, en contradiction avec ses principes fondateurs de solidarité, de gestion paritaire et de progrès continu. Tel est le sens de cette question préalable. Le journal ne pouvait cacher sa joie en sous-titrant le mardi 31 octobre : « Le transfert des cotisations sociales vers la CSG constitue une des réformes clefs de l'exécutif. » De manière « emblématique » en effet, il n'y aura plus en 2019 de cotisation « employeur » au niveau du SMIC. Or la cotisation sociale est un prélèvement sur les profits des entreprises qui ouvre des droits salariaux sur la santé, les retraites, la politique familiale- et j'en passe que les représentants des salariés ont toute légitimité à cogérer. Il n'en est plus de même avec la fiscalisation massive des recettes de la sécurité sociale. Derrière l'écran de fumée de la « hausse du pouvoir d'achat », c'est donc le détournement du salaire indirect, c'est-à-dire des cotisations, qui est organisé. Ainsi, entre 1990 et 2018,

Or la CSG est acquittée à près de 90 % par les salariés et les retraités quand les cotisations sociales sont à 70 % à la charge de l'employeur. Parallèlement, et non sans lien, les dividendes versés aux actionnaires sont passés de l'équivalent de dix jours de salaire voilà trente ans à

Vous vous donnez en réalité les pouvoirs pour imposer au régime le passage progressif d'un droit du salarié généré par la cotisation, particulièrement précieux dans une France à 6 millions de chômeurs, à une prestation sociale uniforme- pourquoi pas ? -, dont vous fixerez- pourquoi pas ? -le montant. La fiscalisation massive du financement de la sécurité sociale, c'est aussi le détricotage

de loi de financement de la sécurité sociale constitue donc un véritable déni de réalité, alors que les hôpitaux publics, les équipes médicales et de soignants, les patients sont déjà au bord de la crise de nerfs. Le plafonnement des dépenses d'assurance maladie à seulement 2 %, si l'on ne prend pas en compte l'augmentation du forfait hospitalier de 18 euros à 20 euros par jour, est insupportable quand les besoins évoluent naturellement de 4,5 Ce sont aussi 10 % des recettes nouvelles déjà insuffisantes qui seront financées par une ponction supplémentaire sur les plus pauvres- assurés sans couverture, handicapés en maison d'accueil spécialisé -, mais aussi sur l'ensemble des patients, l'augmentation quasi inévitable des « mutuelles ». Le développement de l'ambulatoire, dont le bilan réel reste à faire en termes de qualité de prise en charge des malades et des coûts liés aux réadmissions, ne saurait justifier ce nouveau « délitement » de l'hôpital public Je sais bien que le président Macron est passé maître dans les tours de passe-passe, afin de présenter aux Français des reculs comme des avancées. Il faut reconnaître que vous savez aussi jouer de la division pour mieux imposer cette logique libérale, c'est-à-dire l'affaiblissement généralisé de notre système de protection sociale au nom de la sacro-sainte

331 euros pour les moins de 65 ans, seront taxés d'un nouveau prélèvement direct sur leur revenu et leur pouvoir d'achat. Comme si on était riche avec un tel niveau de ressources, que l'on soit d'ailleurs retraité ou salarié En somme, votre conception de la politique sociale, c'est l'alignement vers le bas des revenus modestes. C'est d'ailleurs ce qu'a très bien expliqué le rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, en pointant le fait que les retraités avaient été « moins impactés » par la crise ! En réalité, vous ne digérez pas le fait que la pension moyenne des retraités soit passée de 62,7 % à 66,1 66,1 % du revenu d'activité moyen, ce qui n'est pourtant que la conséquence d'une plus grande activité des femmes notamment. Il est vrai que c'est tout notre système de retraites que vous voulez bousculer en proposant, dès le printemps prochain, une retraite par points, où le montant des pensions pourrait varier à la baisse pour sanctuariser- c'est là le fond -les cotisations patronales à leur niveau le plus bas possible. Ce qui est en train de se passer au niveau des retraites complémentaires en est la parfaite préfiguration. La politique familiale sera aussi une des grandes perdantes de ce budget. Non seulement vous réaliserez une économie de 760 millions d'euros, malgré l'excédent de la branche, mais les quelques mesures positives ne pourront pas masquer le véritable changement de paradigme que vous vous vantez d'imposer à la branche, contre l'avis majoritaire de son conseil d'administration. Ce dernier, en ne vous suivant pas, a marqué à juste titre son attachement à une véritable politique familiale favorisant- je rappelle ce qu'est une politique familiale familiale ! -la natalité, l'autonomie et l'émancipation de la femme et l'épanouissement de chaque enfant. Mais alors que ces indicateurs de la politique familiale sont au rouge, vous accélérez au contraire la fuite en avant de la mise sous conditions de ressources de certaines prestations à un plafond de ressources toujours plus bas. Où est la justice sociale ? Où est la politique familiale, quand les familles exclues de la prestation d'accueil du jeune enfant passeront de 20 % à 30 % des potentielles éligibles ? Les Français doivent savoir, par exemple, que les parents bénéficiaires actuels de la prestation à taux plein gagnant chacun plus de 1 660 euros et accueillant un deuxième enfant en perdront la moitié à partir du 1 avril 2018 Fondamentalement, les difficultés dans l'accès aux soins, la remise en cause de la politique familiale, le matraquage des retraités, l'étatisation de la sécurité sociale ou l'absence

de la prédation toujours plus sauvage des richesses par les privilégiés de l'argent. Faut-il rappeler ici que la fortune des 500 Français les plus riches a été multipliée par sept en vingt ans et que chacun des 100 Français les plus riches

qui n'a jamais été aussi riche, pour donner une autre ambition que l'austérité et la confiscation toujours plus grande des moyens de gestion de la sécurité sociale aux assurés eux-mêmes. Il faudrait au contraire mobiliser les intelligences et les moyens, rassembler les efforts pour lutter efficacement contre la désertification médicale ou le renoncement aux soins, particulièrement problématique dans certains territoires et chez les jeunes par exemple, pour reconstruire un système de prévention en milieu scolaire et au travail en en faisant une vraie priorité nationale et pour mettre fin à la casse

à la Commission européenne dans sa logique austéritaire. Vous imposez, avec le projet de loi de programmation des finances publiques que vous venez de faire voter ces jours-ci, un carcan limitant la croissance des dépenses de santé à 2,3 % sur la période 2018-2022 quand les réponses

que votre attachement aux fondements humanistes de la sécurité sociale

Le scrutin est ouvert.

vous connaissez tous, comme moi, la situation « réelle » des comptes de la sécurité sociale. Malgré une amélioration sensible de la situation financière de l'ensemble des branches, la dette sociale de la France demeure à un niveau très élevé, trop élevé, aux alentours de 5 milliards d'euros cette année encore. Selon la Cour des comptes, le retour à l'équilibre ne pourrait pas intervenir avant 2020. C'est dire l'illusion entretenue jusqu'ici ... Nous sommes réunis aujourd'hui pour entamer l'examen du projet de loi de financement de Il a pour objectif la réduction du déficit de la sécurité sociale à 2,2 milliards d'euros. Madame la ministre, engagés sur le thème de la réduction des dépenses et le retour à l'équilibre, nous ne pouvons que soutenir votre volonté affirmée de réduire ce déficit, à l'impérieuse ce déficit, à l'impérieuse condition, bien entendu, que les mots rencontrent les actes, car un retour à l'équilibre est absolument nécessaire, et pas seulement dans le domaine de la santé C'est sur le volet « santé » que je souhaite intervenir plus particulièrement. Convaincue que la prévention et l'innovation sont les deux piliers d'une gestion moderne et équilibrée des comptes en matière de santé, j'aimerais tout d'abord insister sur les mesures qui leur sont consacrées dans le projet Vous indiquez, madame la ministre, que la prévention sera un axe central de la nouvelle stratégie nationale de santé et qu'elle sera arrêtée d'ici à la fin de l'année. D'ici là, l'une des mesures phares est l'extension d'obligation de vaccination pour les enfants, que je soutiens sans aucune réserve en tant que médecin. C'est nécessaire compte tenu de la grande défiance des Français à l'égard de la vaccination, qui fait courir le risque d'un recul de la couverture vaccinale, avec comme conséquence la réapparition de maladies disparues aux conséquences graves, voire mortelles, pour nos enfants. J'ajouterai même qu'un débat devrait être lancé sur la généralisation de la vaccination contre la grippe des professionnels de santé ; c'est aussi une question d'exemplarité et de solidarité. Il en est de même pour le vaccin contre le papillomavirus. Madame la ministre, mes chers collègues, le constat est préoccupant. Notre pays accuse un retard considérable qui doit nous alerter : seulement 15 % des adolescentes françaises sont vaccinées, contre 90 % en Finlande et 85 % au Royaume-Uni. Nous sommes bien loin des objectifs de 60 % fixés par le plan Cancer 2014-2019.

portugaises, finlandaises ou anglaises, alors qu'il est aujourd'hui considéré comme largement évitable grâce à la vaccination et au dépistage. Je le sais, dans le domaine vaccinal, il vous faut combattre la désinformation, voire parfois l'obscurantisme, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de la situation. Dans ce combat, je serai à vos côtés. Toujours dans le champ de la prévention, j'aimerais évoquer le prix du tabac. Le Gouvernement prévoit plusieurs hausses successives jusqu'en 2020. Le tabac, dont nous connaissons tous les conséquences néfastes sur la santé, doit faire l'objet d'une lutte sans merci de la part des pouvoirs publics, y compris avec le concours de nouvelles formes de communication, parfois innovantes, tout simplement pour atteindre en premier lieu le public jeune.

Je pense notamment aux habitants des territoires frontaliers, comme dans le Grand Est- région où je suis élue -, qui n'hésitent pas à se rendre au Luxembourg, à quelques kilomètres, pour s'approvisionner.

la sécurité sociale, vous avez indiqué qu'en parallèle à la hausse du prix du tabac sera engagée une politique de prévention et de sensibilisation, ainsi que des actions visant à lutter contre la contrebande et à limiter les achats transfrontaliers. le crois, de beaucoup de mes collègues, je souhaite que de telles mesures soient mises en place le plus rapidement possible. Je suivrai avec beaucoup d'intérêt les annonces sur le sujet. Certaines d'entre elles devront nécessairement être portées à l'échelon européen. La prévention, c'est également la généralisation du sport à des fins de santé. L'élaboration d'un plan sport-santé fait partie des mesures annoncées que je soutiens. J'y vois toutefois des contradictions

De plus, je ne vois toujours pas de grande évolution dans le domaine du sport-santé sur ordonnance depuis la publication du décret du 30 novembre 2016, qui permet aux médecins généralistes de prescrire une activité physique. Madame la ministre, quels financements envisagez-vous pour que cette mesure atteigne enfin son objectif ?

En plus d'être inefficace, une telle mesure me semble injuste, car elle touchera prioritairement le porte-monnaie des publics parmi les plus défavorisés et les plus éloignés de la prévention. Encore une fois, l'effort doit être porté sur l'éducation à la santé, qui se révèle bien plus efficace : plus de prévention, c'est moins de maladies chroniques et moins de soins. Encore faut-il avec audace inverser le logiciel, changer les comportements en profondeur dès le plus jeune âge, être ambitieux et innovants et octroyer à la prévention et à l'éducation un budget à la hauteur de l'enjeu L'innovation vient compléter le travail de prévention que je viens d'évoquer. L'article 36 donne un cadre à la généralisation de la télémédecine en permettant notamment la tarification à l'acte. Je salue cette mesure attendue, qui répond à un réel besoin de la médecine moderne. Certes, elle répond aussi en partie aux problématiques des zones de désertification médicale, mais elle doit surtout être appréhendée comme un vecteur d'innovation et accompagner les nouvelles pratiques en matière de santé. Le champ de la formation dans ce domaine devra également appréhender rapidement les nouvelles orientations pour qu'elles soient efficaces sur le terrain.

Dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, les projections à cinq ans indiquent qu'il n'y aura plus qu'un seul médecin généraliste dans une commune de 10 000 habitants que je connais bien. Je ne crois aucunement aux mesures coercitives. vous avez annoncé vouloir doubler les maisons de santé pluriprofessionnelles, les MSP. Cela sera possible si les contraintes sont allégées. À ce jour, il faut environ cinq années pour qu'un projet de MSP aboutisse. C'est beaucoup trop long ; sur les territoires, l'urgence, c'est vraiment aujourd'hui Je crois que, dans ce domaine, il faut faire confiance et accompagner avec souplesse et réactivité toutes les initiatives des acteurs de terrain. C'est aussi cela, la nouvelle forme d'innovation ! Vous avez indiqué vouloir encourager l'expérimentation et son déploiement.

Constatant le phénomène croissant de désertification médicale, les deux praticiens ont décidé de créer une société d'exercice libéral multisite, permettant d'installer des points de consultation de médecine générale sur des territoires considérés comme prioritaires.

comme vous l'avez déclaré dans vos propos, libérez l'initiative ! Libérez-nous d'organisations parfois inadaptées à ce siècle, parfois inadaptées à la révolution numérique en cours, à l'évolution rapide de la société ! Levez les nombreux obstacles bureaucratiques que les professionnels rencontrent. Permettez l'expérimentation, et n'hésitez pas à encourager tout ce qui pourrait être le fruit de l'imagination ou de la créativité dans le domaine de la santé. Le groupe du RDSE se montrera particulièrement attentif au débat, auquel il contribuera de manière positive, afin d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens dans le domaine de la santé. Nous serons particulièrement attentifs au sort réservé à nos amendements. La parole est

disons-le clairement : on peut fustiger à l'infini la hausse de la CSG, l'alignement des plafonds des allocations familiales concernant l'allocation de base de la PAJE sur celui du complément familial, la baisse du coût du travail, qui favoriserait uniquement le patronat, mais on ne peut vouloir à la fois la réduction des dépenses publiques et exiger le maintien des financements actuels d'un certain nombre de prestations. Le Gouvernement veut non pas les abolir, mais en réduire le coût pour avoir un budget conforme aux critères de Maastricht, idée que l'on peut bien évidemment ne pas partager, surtout si l'on se moque des déficits et de la dette. Le budget, la santé, l'assurance vieillesse ... Voilà bien des sujets d'une extrême importance, qu'il conviendrait d'aborder avec le plus grand sérieux et la meilleure projection à long terme si nous voulons que notre système non pas simplement survive, mais puisse être aussi bénéfique et protecteur pour les générations à venir. J'ai souvent évoqué l'introduction d'une pluriannualité dans notre processus budgétaire. Je me réjouis aujourd'hui de voir que ce budget s'annonce dans une vision à long terme et coordonnée des finances de la nation. Le projet que le Gouvernement nous présente ici dans sa philosophie générale a un objectif clair de retour à l'équilibre des comptes pour les années à venir, en s'occupant à la fois des déficits et de la dette, qui devrait être résorbée en 2024. Je souhaite souligner que ce budget s'est construit autour d'une prévision de croissance de 1,7 %, hypothèse semblable à celle de l'OCDE le Haut Conseil des finances publiques a salué la prise en compte d'un scénario macroéconomique à la fois prudent et raisonnable afin de déboucher sur un budget sincère. La part du PIB consacrée aux dépenses de santé dans le monde est en moyenne de 9,92 % selon la Banque mondiale- ce sont les chiffres de 2014. La France dépense de manière assez stable environ 12 % de son PIB, là où les États-Unis y consacrent 17,1 %, chiffre en hausse depuis 1995. Notre pays est souvent pointé comme ayant un bon système, issu des idées généreuses du Conseil national de la Résistance. Mais depuis les Trente Glorieuses, le monde a changé, ne serait-ce que par l'augmentation des dépenses consacrées à la santé- elles sont passées de 6 % dans les années 1960 à 12 % actuellement -et par la baisse du nombre de cotisants depuis le retour des crises économiques successives. Il faudra du courage pour aborder la problématique d'un cinquième sujet, que je ne saurais qualifier de risque, la dépendance. Cet aspect ne peut seulement représenter une variable d'ajustement dans notre système de protection sociale ; il représente un véritable défi

Longtemps négligée, la prévention apparaît essentielle dans la réduction de l'occurrence et de la gravité des pathologies. Avec l'éducation à la santé, le dépistage est un levier essentiel pour notre politique de santé publique. Le texte qui nous est présenté contient deux mesures majeures dans cette lignée. Tout d'abord, l'extension de l'obligation vaccinale à onze vaccins. N'en déplaise aux vendeurs de peur, cette mesure est une bonne mesure.

Les vaccins ont démontré leur efficacité et le rapport bénéfice-risque est nettement en leur faveur. Comment accepter que l'on puisse aujourd'hui mourir d'une maladie qu'un vaccin peut éviter : rougeole, méningite, cancer du foie causé par l'hépatite B ? Dépassons les polémiques sur les adjuvants, puisque d'importants progrès ont été faits sur la tolérance vaccinale, ou sur les bénéfices des laboratoires pharmaceutiques, qui participent eux aussi activement à la recherche. Vient ensuite l'augmentation du prix du tabac. Rappelons que le tabac est la première cause de mortalité en France, cancers et maladies cardiovasculaires confondus. Notre pays est, hélas ! un des champions du tabagisme en Europe. Une fiscalisation plus importante du tabac a fait ses preuves, comme l'a montré une étude australienne, mais il faudra aussi s'attarder sur les effets pervers de cette mesure, qu'il s'agisse de la fraude ou de la contrebande, et développer activement une communication pour pointer les méfaits du tabagisme, en particulier chez les jeunes. J'évoquerai maintenant la question de l'innovation développée par le PLFSS. Il s'agit tout d'abord de l'innovation technologique, que ce soit en matière de diagnostic et de thérapeutique. La recherche, en particulier sur l'épigénétique, discipline de la biologie qui étudie les mécanismes moléculaires modulant l'expression du patrimoine génétique en fonction du contexte, a révolutionné le pronostic de certaines maladies qui, naguère fatales, sont devenues aujourd'hui curables. Certes, ces progrès ont un coût considérable, et il nous faudra réfléchir de façon approfondie à la question du prix du médicament, notamment à l'échelon européen. Bien sûr cette innovation doit bénéficier à tous les patients, mais sans doute devrons-nous faire des choix, y compris sur le reste à charge des pathologies courantes.

Pour clôturer ce court chapitre sur l'innovation, je rappellerai que l'innovation scientifique doit s'accompagner d'innovation éthique, comme le souligne Emmanuel Hirsch dans une récente tribune. La révision des lois de bioéthique en 2018 abordera ce sujet. Comme l'écrivait déjà Rabelais, « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ».

Une réflexion sera menée sur de nouveaux parcours de soins- décloisonnement ville-hôpital -et sur de nouveaux modes de rémunération, tels que la rémunération forfaitaire. En particulier, la tarification à l'acte à l'hôpital, la fameuse T2A, a révélé des effets pervers ; sans doute faudra-t-il remettre ce sujet à plat.

dans sa dimension d'innovation tant scientifique qu'organisationnelle et il n'a d'autre but que de maintenir un système de santé juste, équitable et solidaire, en particulier d'un point de vue générationnel afin de ne pas faire supporter la dette aux générations de demain. Madame la ministre, vous êtes condamnée à réussir : nous vous y aiderons ! La parole est à Mme Laurence Cohen.

Alors que nous examinons ce budget de la sécurité sociale, comment ne pas avoir une pensée pour ce grand humaniste qui fut sénateur, député, maire d'Aubervilliers et ministre de la santé, et qui plaçait l'être humain au coeur des politiques à mener ? J'espère qu'il inspirera nos travaux.

sociale pour 2018 remet en cause les principes fondateurs de la sécurité sociale qui veulent que chacun cotise selon ses moyens et reçoive selon ses besoins. Réduire les cotisations sociales, pour les supprimer, sous prétexte d'augmenter le salaire direct est un leurre, voire une escroquerie intellectuelle. Non seulement c'est une façon d'exonérer le patronat de toute augmentation de salaire, mais c'est couper les vivres à notre système de protection sociale, qui permet à chacune et à chacun de faire face, à égalité, à la maladie, aux accidents du travail, aux besoins de base de la famille et à la vieillesse. C'est faire voler en éclats le principe de solidarité entre générations, entre bien portants et malades, entre actifs et inactifs.

Ainsi, les plus riches disposeront d'une assurance privée protectrice et la majorité des Français d'une assurance minimaliste. Comment ne pas dénoncer les budgets des PLFSS successifs qui contraignent les dépenses de santé, à la fois au détriment de l'offre et de la qualité des soins, mais aussi des conditions de travail des personnels ? Vous nous dites, madame la ministre, que 30 % des dépenses de santé ne seraient pas pertinentes. Ainsi, les Françaises et les Français dépenseraient trop pour se soigner ! Faut-il rappeler qu'en France les dépenses de santé s'élèvent à 11 % des richesses

Parmi vos propositions de financement, il y a l'augmentation de la CSG. Quoi de plus injuste quand on sait qu'elle repose à 70 % sur les revenus du travail et à 18 % sur les retraites ? sur les retraites ? Quoi de plus injuste quand on sait que 2,5 millions de retraités modestes ne bénéficieront pas des compensations financières du Gouvernement ? Quoi de plus injuste quand on sait que cette cotisation entre pour partie dans le revenu imposable ? Ainsi, vous supprimez l'impôt sur la fortune pour les cent foyers les plus riches tandis que vous demandez toujours plus aux autres. Nous ne voterons bien évidemment pas cette hausse de la CSG ! Nous ne sommes pas face à des choix de bons gestionnaires visant à réduire des dépenses inutiles, mais nous sommes face à des choix de réduction drastique du périmètre de la protection sociale et du service public de santé : nous sommes face à des choix de société Toujours au nom des 30 % des dépenses de l'assurance maladie non pertinentes, vous justifiez un ONDAM à 2,3 % alors que, selon la Confédération des syndicats médicaux français, la croissance naturelle des dépenses est de 4,5 %. Sur les 4,2 milliards de restrictions budgétaires pour la branche maladie, l'hôpital public devra supporter 1,2 milliard de coupes sombres. Comment résister à cette nouvelle ponction après les cures d'austérité successives qu'il a subies avec Mmes Bachelot et Touraine ? Comment pouvez-vous affirmer vouloir recentrer l'hôpital sur l'excellence et la haute technicité quand vos choix budgétaires vont entraîner de nouvelles fermetures de lits, la disparition de services et d'hôpitaux, alors que les urgences sont ultra-saturées, que les déserts médicaux gagnent du terrain et que les personnels sont à bout ? Comment prétendez-vous parfaire l'ambulatoire dans un tel contexte avec des manques de généralistes, de spécialistes, de personnels paramédicaux, avec des centres de santé en nombre insuffisant ? Permettez-moi, à cet instant, de rendre hommage au personnel hospitalier mobilisé il y a deux ans à l'occasion des attentats. Ce sont les mêmes agents dévoués au quotidien pour l'intérêt général qui permettent à l'hôpital de tenir debout alors que leurs moyens sont réduits chaque année.

Il n'y a pas besoin d'avoir travaillé vingt-cinq ans à l'hôpital, madame la ministre, pour se rendre compte de la dégradation des conditions de travail du personnel hospitalier et de la détérioration de la qualité des soins. La semaine dernière, un neurochirurgien a mis fin à ses jours au CHU de Grenoble : le syndrome France Télécom atteint, hélas ! l'hôpital. Il faut d'autres choix que ce sous-financement chronique des hôpitaux, cette gestion purement comptable et ce management qui met les soignants en souffrance. Les personnels se mobilisent d'ailleurs un peu partout

Alors que, selon le dernier baromètre Secours populaire français-IPSOS, quatre Français sur dix renoncent à se soigner du fait de l'augmentation incessante du reste à charge, le forfait hospitalier va augmenter

Que dire de la transformation du CICE en exonération pérenne des cotisations sociales pour les salaires en dessous du SMIC ? Contrairement aux éléments de langage du Gouvernement, le CICE n'est pas supprimé. Au contraire, il est sanctuarisé jusqu'en 2019 avant la disparition définitive des cotisations à la branche famille, soit 25 milliards d'euros en moins pour les comptes de la sécurité sociale. Comment admettre qu'aucun bilan ne soit tiré de ce CICE ? Ce sont 45 milliards de deniers publics, de 2013 à 2015, qui ont servi à la création de seulement 100 000 emplois : beaucoup d'argent pour un bien piètre résultat

Aujourd'hui, tel un illusionniste, le Gouvernement communique sur l'augmentation de 30 % du montant du complément de garde pour les familles monoparentales. Mais derrière ce rideau de fumée, l'allocation de base de la PAJE est réduite pour tout le monde. la CNAF, 44 000 familles obtiendront un gain mensuel moyen de 70 euros par enfant gardé, tandis que la baisse du montant de la PAJE entraînera une perte de 500 euros sur la durée de versement de la prestation les familles les plus modestes et de 250 euros pour les familles de catégorie intermédiaire ayant de jeunes enfants. À cette diminution du montant, s'ajoute la baisse du plafond de la prestation, ce qui exclura demain près de 10 % des familles qui pourraient percevoir aujourd'hui En réalité, le Gouvernement veut transformer la branche famille universelle en un système d'aide ciblée vers les ménages les plus précaires. C'est l'amplification de la rupture de l'universalité des allocations familiales déjà assumée durant le précédent quinquennat. Ce double discours se retrouve à propos de la revalorisation de 100 euros du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, alors que le recul de la date de revalorisation au 1 janvier 2019 rapportera 380 millions d'euros en 2018 au budget de l'État. L'adaptation de la société au vieillissement est un véritable enjeu pour notre modèle de protection sociale, comme l'a souligné Dominique Watrin. Plutôt que de considérer les retraités uniquement comme des personnes exploitables à volonté ou d'envisager de moduler moduler le montant des pensions avec votre projet de réforme des retraites, il serait temps d'investir massivement pour améliorer les conditions de travail du personnel d'aide à domicile, des aidants familiaux et du personnel travaillant dans les établissements qui subissent la réforme de la tarification. En aucun cas ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ne règle ces problèmes. Ajoutons à cela la suppression du RSI, du tiers payant généralisé et le passage de trois à onze vaccins obligatoires. Si nous soutenons les vaccins, en général, en tant que formidables protections pour les populations, nous demandons des garanties pour une sécurité vaccinale, notamment en ce qui concerne les adjuvants. L'absence de transparence a créé de la défiance et ce n'est pas en imposant les vaccins que la confiance va revenir. Il est troublant de constater que vous suivez les directives de grands laboratoires pharmaceutiques qui déclaraient ne pas pouvoir sortir trois vaccins- le DT-Polio -, mais qui aujourd'hui en sortent onze ! Il faut dire que le rapport financier est nettement plus avantageux pour eux : trois vaccins étaient facturés un peu plus de 20 euros en 2008 tandis qu'ils pourront aujourd'hui empocher 350 euros pour onze vaccins Si la mesure devient obligatoire, elle doit être totalement gratuite et prise en charge par la sécurité sociale. Il faut aller au bout de cette logique, madame la ministre, c'est le sens d'un amendement que nous défendrons Plus de moyens pour l'hôpital public et la médecine de ville, c'est possible : il suffit d'en avoir la volonté politique. Pourquoi n'avoir rien prévu contre la fraude patronale, qui coûte la bagatelle de 20 milliards d'euros par an aux comptes de la sécurité sociale selon la Cour des comptes ? Vous êtes, à juste titre, attentive à l'argent public, Pourquoi ne pas faire respecter la loi par les entreprises qui ne l'appliquent pas concernant l'égalité salariale ? La Fondation Concorde a estimé le manque à gagner pour l'économie française à 62 milliards d'euros et à 25 milliards d'euros de cotisations pour la sécurité sociale. Pourquoi ne pas décider la suppression de la taxe sur les salaires à l'hôpital, qui rapporterait 4 milliards d'euros, alors que votre gouvernement n'hésite pas à dilapider 3,4 milliards d'euros de deniers publics en supprimant l'ISF ? De l'argent, il y en a supprimer les exonérations de cotisations patronales pour les entreprises qui ne créent aucun emploi en contrepartie, ce sont 45 milliards d'euros par an, soit 10 % de la totalité du budget de la sécurité sociale Être en prise avec les évolutions de son temps, c'est défendre un système de protection sociale juste, solidaire et pérenne qui prend ses racines dans les conquêtes du Conseil national de la Résistance, sous l'impulsion d'Ambroise Croizat. C'est défendre les principes fondateurs de la sécurité sociale tout en étant favorables à son évolution. C'est l'ambition que je porte avec mon groupe, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Nous voulons une évolution qui aille vers une plus grande prise en charge des soins, qui laisse moins de place aux complémentaires santé, et non l'inverse comme vous le proposez. Au XXI siècle, dans un pays riche comme la France, il est possible que la sécurité sociale rembourse les soins à 100 %, y compris les soins optiques, dentaires et les prothèses auditives. Il est possible de mener une politique ambitieuse de prévention qui passe notamment par l'arrêt du démantèlement de la médecine scolaire et de la médecine du travail, conditions de travail, les CHSCT, dans la réforme du code du travail. Il est possible de développer l'innovation, d'améliorer la sécurité sanitaire par la création d'un pôle public du médicament et de la recherche.

en tenant compte de la politique salariale, environnementale des entreprises, mais également en supprimant les exonérations de cotisations patronales en tout genre. Les difficultés de la sécurité sociale sont organisées volontairement sous la pression de ceux qui possèdent les richesses et qui se font sans cesse exonérer de leur contribution au bien commun. Notre groupe ne peut entériner un tel projet de démantèlement démantèlement de notre système de protection sociale, contraire à l'intérêt du plus grand nombre. C'est pourquoi nous voterons contre ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, à moins que nos amendements soient pris en compte. On peut toujours rêver

était attendu. Quelle vision d'une sécurité sociale du XXI siècle ? Quelles réponses apportées aux défis de notre système de santé : allongement de la vie, polypathologies, maladies chroniques, innovations médicamenteuses, inégalités territoriales et financières d'accès aux soins, culture de la prévention- national du cancer, pourraient être évités par des mesures alimentaires, comportementales et d'hygiène de vie -, soins dans la durée exigeant des interventions combinées de professionnels de santé Une considération doit primer toutes les autres : la dimension humaine. Tel est l'héritage des ordonnances d'octobre 1945, le coeur de notre vivre ensemble, avons la responsabilité de maintenir les fondements de solidarité en leur donnant une efficience dans la réalité d'un monde ouvert à toutes les compétitions et où l'individualisme triomphe.

La pérennité de notre sécurité sociale repose sur notre responsabilité collective, celle des professionnels, celle des patients, des élus, à retrouver un équilibre financier, condition de la confiance de nos concitoyens en l'avenir, mais aussi enjeu de dignité et de responsabilité envers nos enfants et petits-enfants. La sécurité sociale était excédentaire en 2001.

l'écart entre la hausse de la CSG dès le 1 janvier prochain et les baisses de cotisations chômage et maladie ? Madame la ministre, du doute naît la suspicion : pouvez-vous nous éclairer précisément sur ce point ?

à la condition, non satisfaite à ce jour, d'excédents à venir des branches ou de recettes nouvelles qui permettraient de couvrir 20 milliards d'euros de déficits cumulés de l'ACOSS. Prenons garde à la dangereuse illusion entretenue par les taux d'intérêt faibles ou même négatifs sur le court terme. Madame la ministre, nous serons à vos côtés quand vous affirmerez la prévention, premier objectif de la stratégie nationale de santé. L'article 11 porte l'obligation vaccinale à onze vaccins pour les enfants de moins de 24 mois. Quand une enquête réalisée dans soixante-sept pays en octobre 2016 classe la France championne du monde de la défiance vaccinale, quand des enfants meurent de la rougeole dans notre pays, il est rassurant que l'État prenne ses responsabilités. L'urgence sanitaire impose l'obligation. En ce mois de novembre sans tabac, créé sur l'initiative de Marisol Touraine en 2016, une nouvelle étape est engagée dans la lutte contre la consommation du tabac, avec l'objectif d'un paquet de cigarettes à 10 euros en 2020. Les prix de vente sont fixés par les fabricants ; je reviendrai dans le cours du débat sur les modalités retenues. J'insiste sur trois points : l'accompagnement par des actions de communication en direction des jeunes avec leur langage, leurs codes ; l'évolution de la profession de buraliste qui structure nos territoires ; l'urgence, que vous avez évoquée tout à l'heure, de la lutte contre le commerce illicite de tabac en France, le plus important d'Europe, avec près de 9 milliards de cigarettes par an.

que la disposition « vise non pas à gagner de l'argent sur la vente des boissons sucrées, mais à inciter les industriels à mettre moins de sucre dans les boissons ». Or il semble que les valeurs adoptées

La CSG, créée par Michel Rocard, s'est appliquée au taux de 1,1 % pour la première fois en 1991. Augmentée par les gouvernements Balladur, puis Juppé, devenue pour partie déductible, elle progressera en 1999 de 4,1 points sous le gouvernement Jospin en contrepartie d'une baisse de 4,75 points des cotisations maladie, mais à l'époque la hausse limitée à 2,8 points pour les retraités était compensée totalement. L'idée était déjà de rendre du pouvoir d'achat aux aux salariés. Vous n'êtes pas dans cette continuité, vous n'y êtes pas en raison du transfert assumé entre les générations. Une redistribution des ménages de plus de 60 ans vers les ménages de moins de 60 ans est-elle juste ?

quand dans le même temps la suppression d'une partie de l'ISF et la mise en place de la allégeront de plusieurs milliards d'euros la contribution à la solidarité nationale des familles les plus aisées. Nous présenterons un amendement visant à supprimer cette disposition. Nous soutiendrons de même un amendement de suppression de l'alinéa 6 de l'article 44. Madame la ministre, vous avez tort de supprimer le caractère obligatoire du tiers payant, qui va dans le sens de l'histoire. C'est un marqueur social répondant à une des difficultés d'accès aux soins. Le rapport de l'IGAS est nuancé. Il sépare la part sécurité sociale de la part des complémentaires. La mise en place est techniquement réalisable à brève échéance pour la part sécurité sociale- 16,50 euros sur une consultation de 25 euros. Or, après la décision du Conseil constitutionnel, constitutionnel, seule cette part pouvait voir le tiers payant s'appliquer au 30 novembre. Il était possible d'avancer en deux temps, progressivement, sans bras de fer avec les médecins,

Madame la ministre, pouvez-vous nous préciser le calendrier après la remise du rapport ? Dans la branche maladie, les articles 35 et 36 ouvrent un cadre général pour favoriser les expérimentations en matière d'organisation des soins, pour développer la télémédecine par le financement conventionnel de la téléexpertise et de la téléconsultation. J'en approuve la philosophie, même si des points doivent être précisés ou posent question, comme la composition et le rôle des comités stratégiques et techniques ou le montant alloué au fonds d'innovation. L'enjeu est bien de briser les rigidités, les cloisonnements existants, de remettre en cause le seul paiement à l'acte pour adopter des logiques de parcours ou de séquences de soins, de favoriser l'exercice collectif. Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur le lien- s'il y en a un, ce que je souhaite -des articles 35 et 36 avec les logiques de territoires déjà créées grâce aux équipes de soins primaires et aux communautés professionnelles territoriales de santé ? trois sujets d'inquiétude. Premièrement, l'hôpital public n'assure ses missions que grâce au formidable engagement et au total dévouement du personnel soignant- médecins, personnels paramédicaux -auquel je rends hommage. Quand, chaque année, plus de dix millions de personnes se rendent aux urgences, à l'interface de la médecine et des maux de la société, il y a obligation à redonner du sens à l'hôpital public.

empreint de jugement, il est une véritable violence et entraîne le repli. » Nous sommes au coeur de nos préoccupations pour 2018. La parole

mettre en place, en coconstruction avec les élus, un salariat pour les médecins généralistes qui seraient embauchés par un hôpital ou une clinique et qui pourraient intervenir dans les MSP. Ce modèle semble attractif.

à 70 %. Pour les malades en difficulté financière, il faudrait simplement ajouter dans la loi que le tiers payant doit s'appliquer à la demande du patient. Ce serait très simple

sociale pour 2018 met en place la transformation du CICE et du CITS en allégement des cotisations sociales, à compter du 1 janvier 2019.

sociale traduit une volonté de retour à l'équilibre financier, le choix de privilégier des mesures conjoncturelles a été retenu au détriment de réformes structurelles.

en effet été possible de transférer l'ensemble des déficits de l'ACOSS à la CADES en procédant à une augmentation de la CRDS de 0,25 %, sans toucher à la durée de vie légale de la CADES. C'eût été une démarche vertueuse, permettant de revenir à l'équilibre financier, sans exposer l'ACOSS à la variation des taux d'intérêt, dont on peut craindre qu'elle ne survienne dans les années à venir, tant les marchés financiers sont fébriles. Dans un tel cas de figure,

principaux acteurs de terrain et après une concertation plus que limitée, pourrait être assimilée à un cavalier législatif. Cette

car il marquera la trajectoire que vous comptez donner à votre politique sociale, madame la ministre. Les annonces se sont multipliées ces dernières semaines : stratégie nationale de santé, lutte contre les déserts médicaux, lois de bioéthique, retraites, assurance chômage. C'est l'ensemble de notre politique sociale que vous comptez réformer, en tout début de quinquennat. Nous approuvons la méthode qui consiste à engager une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés avant de faire des propositions. Il n'est plus acceptable que les réformes soient uniquement inventées dans des et traduites dans des cabinets ministériels avant d'être votées en bloc par des majorités aux ordres. Consultez, discutez, inspirez-vous des expérimentations et idées développées dans les territoires de métropole et d'outre-mer. Je m'exprimerai sur les équilibres et les recettes de ce projet de loi de financement de

La protection sociale était réhabilitée, les comptes à l'équilibre, les retraites sauvées, les hôpitaux financés : le satisfecit était total. La majorité sénatoriale avait alors exprimé des réserves- c'est peu dire -quant à la sincérité du texte qui était soumis au Sénat. Votre texte, madame la ministre, le confirme. Le déficit de la branche maladie était beaucoup plus dégradé que ce qui avait été prévu : il est de 4,1 milliards d'euros au lieu des 2,6 milliards d'euros Dindar aura l'occasion de le développer concernant la branche vieillesse : le Gouvernement avait fait preuve d'imagination pour afficher des comptes sous un jour favorable. Le recours à des artifices comptables n'est pas l'apanage de votre prédécesseur il faut le reconnaître, tous les gouvernements y ont recouru. Les lois de financement de la sécurité sociale sont des textes difficiles à appréhender, techniques, où la communication prend logiquement une place importante. J'espère, madame la ministre, que vous assumerez vos projets de loi de

Quant à l'ONDAM, la progression de 2,3 % que vous proposez serait obtenue au prix d'un important niveau d'économies, de près de 4,2 milliards d'euros. Des objectifs exigeants, qui dépendent en partie d'informations tendancielles que nous ne maîtrisons pas.

par la baisse de leurs cotisations sociales, financée par une hausse de la CSG. L'article 7 va très vraisemblablement faire l'objet de nombreuses discussions dans cet hémicycle. Est-il juste de faire supporter cette baisse Est-il juste de faire supporter cette baisse de cotisations par les retraités ? Certes, une partie d'entre eux bénéficiera d'une baisse de la taxe d'habitation, dont l'application, elle, est étalée sur trois années. Certains, cependant, subiront une perte nette de leur pouvoir d'achat. On peut gloser des heures sur les chiffres, trouver les exemples que l'on veut ; à ce jeu chacun développe des trésors d'imagination, tous plus documentés les uns que les autres. Il y a là, en réalité, une question générale, un enjeu de société : doit-on solliciter davantage les retraités, notamment les plus modestes d'entre eux ? Nous aurons l'occasion d'en débattre, et le groupe Union Centriste proposera des solutions alternatives. J'en viens au sujet, ô combien sensible, du RSI. Vivement critiqué pour les erreurs dont les indépendants font les frais dans le calcul de leurs cotisations ou de leur retraite, il a concentré les critiques de la majorité, si ce n'est la totalité, des candidats à la présidence de la République. Emmanuel Macron met donc en oeuvre une promesse de campagne. Il n'en demeure pas moins que des doutes et des inquiétudes subsistent sur les modalités de la réforme

Je terminerai sur les recettes, en abordant brièvement la question de la fiscalité du tabac. La lutte contre le tabagisme est un enjeu crucial de santé publique, et il est démontré que l'augmentation du prix des paquets de cigarettes conduit à une diminution de la consommation, au moins dans un premier temps. Les consommateurs, en effet, se tournent soit vers les revendeurs frontaliers- je puis vous en parler en connaissance de cause, en tant que sénateur mosellan -, soit vers les marchés de contrebande. Augmenter le prix du tabac sans lutter efficacement contre la fraude est donc inutile et n'aura qu'un seul effet : faire disparaître le métier de buraliste. Il faut accentuer la lutte contre la contrebande et veiller à l'uniformisation, à l'échelle européenne, du prix des paquets de cigarettes. Il me semble que vous vous y êtes engagée, madame la ministre.

Vous abordez la question de la prévention principalement l'extension de l'obligation vaccinale. Cette mesure fait partie des choix de société sur lesquels nous devons être particulièrement attentifs. Il existe des doutes, fondés ou non, sur la dangerosité des vaccins ou des adjuvants qu'ils contiennent. Cela ne nécessiterait-il pas un état des lieux plus approfondi ? Je pense, par exemple, à la question de la vaccination des adolescents. Un sujet qui n'apparaît pas, alors qu'il le mériterait, est celui de la médecine scolaire. Médecins et infirmières scolaires sont des rouages essentiels de la prévention. Et pourtant, depuis des années, l'État fait trop peu pour améliorer les conditions de travail de la médecine scolaire, au point que l'Académie de médecine tire la sonnette d'alarme. C'est dans ces services que peuvent être dépistés les grands problèmes de l'adolescence : addictions, obésité, troubles neuropsychiques. Nous soutenons l'article 35 sur la mise en place d'un cadre légal permettant le déploiement d'expérimentations innovantes. Il faut encourager le décloisonnement sur le terrain, dans les départements notamment. Tel devra être le cas en matière de télémédecine, je parle ici de l'article 36 : c'est une des solutions visant à remédier à la désertification médicale. Il est urgent d'agir en la matière. Pour conclure, sachez, madame la ministre, que les sénateurs du groupe Union Centriste abordent l'examen de ce texte de manière tout à fait positive. Nous aurons des discussions,

nous entamons ce jour l'examen du premier projet de loi de financement de la sécurité sociale de ce quinquennat. Même s'il s'agit d'un projet de loi de financement ô combien important, je n'entrerai pas dans le détail de ses équilibres financiers, d'autres orateurs s'étant largement exprimés sur ce sujet.

En tant que professionnelle de santé, je ne peux que me féliciter du contenu de ce PLFSS dans sa partie santé, que ce soit en matière de prévention, de pertinence des soins ou d'innovation. Le nier serait un manque d'honnêteté intellectuelle et contraire à ce que je pense être bon pour la santé de nos concitoyens. Je salue également le financement de plus de 4 500 places d'EHPAD et de 1 500 places d'accueil de jour. C'est une bonne nouvelle pour nos territoires et pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Mais j'appelle votre attention, madame la ministre, sur les choix que vous-même et les agences régionales de santé serez amenés à faire. Dans certains départements, des lits d'EHPAD

Le Gouvernement prétend pouvoir régler ce problème en sollicitant les étudiants en médecine et les médecins retraités. Si la décision de favoriser le cumul emploi-retraite pour les médecins je soutiens l'idée d'exonérer de cotisation vieillesse les médecins pouvant prétendre à une retraite à taux plein, mais qui font le choix, faute de successeur, de prolonger leur exercice en zone sous-dotée. Mais n'est-ce pas insuffisant ? Ne peut-on pas envisager de soigner avec des médecins diplômés et en âge de le faire ? On ne peut pas continuer à utiliser des méthodes de substitution, il est grand temps de réfléchir à des solutions qui permettront l'installation de nouvelles générations de médecins et le développement de délégations de tâches entre professionnels de santé. Les départements se mobilisent pour attirer de nouveaux professionnels de santé ; beaucoup font le choix de l'incitation pour remédier aux départs en retraite de nombreux médecins. Prenons l'exemple de la Charente-Maritime, que je connais bien : ce département propose des bourses d'études aux internes en médecine générale, en contrepartie d'une installation de quatre ans au minimum dans une partie du département de la désertification médicale. Plus au sud, l'Aveyron propose un accompagnement personnalisé des futurs médecins souhaitant s'y installer. La ruralité est dynamique, innovante, mais ces politiques départementales ne peuvent être efficaces si elles ne sont pas accompagnées d'une réforme structurelle de l'organisation de la médecine. La remise à plat du a été une piste longuement évoquée pour faire face à cette situation alarmante. Cette solution a ses adeptes et, surtout, ses opposants, mais force est de constater que, sur trois médecins qui s'installent, un a été diplômé à l'étranger. Aussi, il devient urgent d'innover afin de répondre aux enjeux démographiques. Le Gouvernement entend régler la question des déserts médicaux en construisant des maisons de santé en grand nombre. Ce sont évidemment des équipements de qualité, qui offrent de très bonnes conditions de travail, mais encore faudrait-il qu'il y ait des médecins pour s'y installer ! Le problème majeur des maisons de santé, c'est qu'elles n'ont pas fait neuf ans de médecine et que les murs ne soignent pas La question des déserts médicaux ne peut pas être entièrement réglée par des mesures directement liées à la santé. Ces zones oubliées de la République doivent bénéficier de soutiens supplémentaires de la part de l'État. Tout à fait consciente des attentes des jeunes médecins en termes de qualité de vie personnelle, je pense que l'attractivité de ces territoires passe par la mise en place d'un réseau internet de très haut débit et par le maintien d'un minimum de services publics en zone rurale. C'est une question d'aménagement du territoire- à cet égard, permettez-moi de rappeler que le réseau des officines de pharmacie est exemplaire en matière d'aménagement du territoire national et qu'il constitue une véritable colonne vertébrale en matière d'accès à la santé. Comme le médecin généraliste est la pierre angulaire des soins de ville, l'hôpital est le pilier de notre système de santé, mais il est l'un des grands perdants du PLFSS pour 2018, puisqu'une économie de plus d'un milliard d'euros lui est encore demandée. Les gouvernements successifs des cinq dernières années ont pratiqué la politique du « rabot » sur le dos de l'hôpital. Les conséquences sur la qualité des soins et sur les conditions de travail du personnel hospitalier L'hôpital a su prendre le virage ambulatoire, mais ne perdons pas de vue l'intérêt du patient ni celui du personnel, et ne risquons pas la sortie de route. L'intérêt financier prévaut depuis longtemps par rapport à l'intérêt de santé publique, mais n'avons-nous pas atteint les limites de cette politique ? Nous ne pouvons plus demander encore de telles économies à l'hôpital et à l'industrie pharmaceutique. Le numérique, la télémédecine, avec téléconsultation et téléexpertise, et l'intelligence artificielle sont autant d'outils qu'il faut encore mieux intégrer pour améliorer la prise en charge des patients. Sur cet aspect, vous avez compris les nouveaux enjeux du domaine médical, mais il faudra aller plus loin et plus vite. L'hôpital public exerce d'autres missions. La recherche demeure une priorité, car elle est source d'innovations médicales et pharmaceutiques. La formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers est également l'une des prérogatives de l'hôpital ; cette transmission du savoir est essentielle pour le maintien de la qualité des soins français ; il faut continuer. Si le Gouvernement n'apporte pas de solutions viables au monde hospitalier, alors il doit se résoudre à donner plus d'autonomie aux hôpitaux, à remettre sur un pied d'égalité les cliniques et les hôpitaux en matière de missions de service public. De grâce, essayons, innovons, faisons preuve d'audace ! Il n'y a rien de pire que la résignation et l'attentisme. Parce que le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et l'innovation thérapeutique sont les enjeux d'aujourd'hui et de demain, des réformes structurelles s'imposent. La feuille de soins proposée par le Gouvernement est donc incomplète, trop prudente et parfois inadaptée à la pathologie observée. Les Français sont en droit de réclamer une qualité de soins décente ; les professionnels de santé sont en droit de réclamer des conditions de travail à la hauteur de l'énergie qu'ils dépensent dans l'exercice de leur profession. La tâche est immense et on ne peut plus se permettre d'attendre. Soigner les soignants est notre mission aujourd'hui ; la santé du monde médical est en effet déclinante. En conclusion, parce que le patient doit rester au coeur de nos préoccupations, je citerais le cruciverbiste Serge Mirjean, qui disait : « L'hôpital est un établissement public où les malades ont leurs maux à dire. » Bravo ! La parole

sociale pour 2018 que nous examinons cette semaine, le premier de la nouvelle législature et du quinquennat, cumule à mon sens deux qualités essentielles. il est marqué du sceau de la responsabilité, car il poursuit la trajectoire favorable des comptes sociaux entamée sous le gouvernement précédent. Les chiffres ont été rappelés, le déficit cumulé du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse s'établira en 2018 à 5,2 milliards d'euros, contre 7,8 milliards d'euros L'objectif est d'atteindre l'équilibre d'ici à 2020, et d'apurer la dette de la sécurité sociale d'ici à 2024. Ensuite, ce budget est le fruit de choix assumés et d'une volonté de conduire sans attendre des réformes structurelles importantes pour assurer non seulement la pérennité de notre système de sécurité sociale, mais aussi un meilleur service à ses bénéficiaires. Qu'il s'agisse de la baisse des cotisations des salariés, de la hausse de la CSG, de la transformation du CICE et du CITS en allégements de cotisations patronales, des mesures en faveur des indépendants ou de la politique familiale, il s'agit bien, chaque fois, d'oser faire des choix oser libérer le pouvoir d'achat des actifs, oser augmenter la participation du capital au financement de la protection sociale, oser orienter la politique familiale vers la lutte contre la pauvreté et vers la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Comme l'a indiqué mon collègue Michel Amiel, notre groupe soutiendra donc, dans son ensemble, ce budget équilibré, responsable et réformateur. Permettez-moi de revenir à présent sur quelques mesures de ce PLFSS. qui concerne la prévention en santé, je m'associe pleinement à l'augmentation significative de la fiscalité sur le tabac, donc du prix de celui-ci. Je constate que ce volontarisme fiscal se double d'un engagement à lutter contre les marchés parallèles et à réviser la directive européenne n°

À défaut, toute politique nationale de prévention par le prix manquera sa cible et achèvera de déstabiliser nos buralistes en zone frontalière. Pour ce qui concerne les mesures de couverture vaccinale, je tiens, là encore, madame la ministre, à vous apporter tout mon soutien dans votre volonté de protection générale de la population, mais aussi de cohérence et de lisibilité. En effet,

Or le bénéfice d'une couverture vaccinale accrue contre les maladies graves ne me semble pas discutable. C'est pourquoi je voterai le passage de trois à onze vaccins obligatoires pour qu'un enfant soit accueilli en collectivité. Quant à la télémédecine, l'expérimentation menée dans certains territoires depuis 2009 a permis de tester plusieurs modalités de mise en oeuvre. Dans le Haut-Rhin, une solution innovante de téléconsultation a été développée et expérimentée avec succès pour limiter les effets de la désertification médicale. Aussi, je me réjouis que, dès 2018, la téléconsultation sorte du champ de l'expérimentation pour être généralisée. Pour terminer, je souhaite dire quelques mots du sort de la branche famille au sein du PLFSS. Rappelons que, au total, un effort de 70 millions d'euros est consenti pour la politique familiale en 2018, qui sera une année de transition. Nous reviendrons dans le débat sur certaines mesures. Notre défi premier, collectif, immense, reste celui de la pauvreté des enfants dans notre pays. Malgré de nombreux dispositifs, la situation ne s'améliore pas assez vite ; madame la ministre, personne ne peut s'en satisfaire. Il est en effet grand temps de repenser les objectifs et les mécanismes de notre politique familiale. La simplification du système des prestations familiales est plus qu'un objectif louable, c'est une urgence ! Vous aurez tout mon soutien pour vous attaquer à celle-ci au cours des mois à venir. La parole

Je concentrerai mon propos sur les branches famille et vieillesse, et sur l'accès aux soins, thématiques qui touchent au plus près la vie quotidienne d'un grand nombre de Français. À mon tour, je tiens à saluer le travail de tous nos rapporteurs, qui éclaireront nos débats d'une analyse fine des dispositions que nous examinerons. je veux vous dire, madame la ministre, que vos premiers mois d'action à la tête de ce ministère nous rassurent. Vous agissez avec méthode, en lien avec le terrain, et vous semblez animée de la volonté de trouver des solutions pérennes, loin des dogmes qui provoquent l'immobilisme, voire qui créent de nouvelles difficultés.

Nous serons des alliés et la voix des élus de terrain, celle des collectivités que nous représentons. J'en viens au PLFSS, que nous allons examiner tout au long de la semaine. Concernant la branche famille, je soutiens, ainsi que l'ensemble de mon groupe, la position développée précédemment par la rapporteur Élisabeth Doineau. Les décisions prises par le précédent gouvernement ont ébranlé l'universalité des allocations allocations familiales qui caractérisait la politique familiale depuis des décennies. L'article 26 du PLFSS pour 2018 laisse à penser que vous prenez la même direction, allant ainsi à l'encontre de l'esprit originel des allocations familiales. le regrette, et je soutiendrai la suppression de cet article. La politique familiale n'est pas seulement un acquis historique, elle tient aussi à une vision de la société et à une certaine idée de la France.

Comprenez-le bien, nous serons favorables au versement de la majoration du complément familial pour les familles les plus pauvres et monoparentales- elles sont nombreuses, dans les territoires d'outre-mer comme en France hexagonale

Madame la ministre, mes chers collègues, parler des personnes âgées m'amène à aborder une question transversale, celle de l'accès aux soins pour les plus fragiles de nos concitoyens en perte d'autonomie.

proposé de parvenir en 2022 à l'absence de reste à charge pour les assurés sur les frais d'optiques, de soins dentaires et d'audioprothèses- vous venez de confirmer ce choix et nous saluons ce progrès.

Nous savons également que les personnes âgées s'inquiètent aussi du reste à charge sur tous les autres produits remboursés, qui augmente avec l'âge, puisque le coût des mutuelles augmente à partir de 60 ans pour les personnes en perte d'autonomie. Le dossier de l'accès aux soins exige donc une réforme harmonisée, simplifiée et des offres labellisées plus justes, à mesure que croît la perte d'autonomie. Les personnes porteuses de handicap sont également concernées par ces dispositifs d'accès aux soins et à la santé.

Ces réformes doivent être conduites sans s'exonérer d'une vision globale des enjeux et des modalités de la politique familiale, et je sais que c'est l'esprit de ce gouvernement, qui sera sensible au pragmatisme des élus locaux, principalement de ceux qui sont chargés, dans les départements, des personnes âgées et des publics vulnérables dans les départements. Le débat parlementaire doit aussi bénéficier de cette simplification. En tant que nouvelle sénatrice, sénatrice, j'aurais aimé aborder l'ensemble de la politique sociale cette semaine, sans attendre le projet de loi de finances, et parler de l'AAH, des personnes porteuses de handicap et des sujets que je viens d'évoquer, qui sont intimement liés. Or nous travaillons dans deux cadres financiers différents. Comme vous le dites, la politique de la famille doit évoluer comme la famille évolue, mais il me semble important que toutes les familles y aient accès. Je ne pourrais pas terminer mon propos sans vous faire voyager un peu, de Mayotte à La Réunion, de la Guyane aux Antilles, sans oublier Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Papeete, ni, bien entendu, Wallis-et-Futuna.

du quinquennat avec bienveillance, mais une bienveillance qui ne nous empêchera pas de nous opposer à certaines mesures lorsque nous estimerons qu'elles ne prennent pas une direction satisfaisante, celle du redressement de nos comptes sociaux au profit d'une meilleure protection pour tous.

du développement des pathologies chroniques, de la dépendance, de l'intrication du médical et du social et de la place des facteurs environnementaux. Il importe que le rôle des différents acteurs du système de soins, leurs missions, leurs modes d'organisation et leur coordination répondent bien à ces enjeux et ne restent pas figés dans des représentations passées. passées. L'hôpital d'aujourd'hui et de demain n'est bien sûr plus celui de 1958, ni même celui de 2007. Or les moyens qui lui sont accordés ne lui suffisent clairement plus pour assurer ses missions actuelles.

Les investissements nécessités par le développement de l'ambulatoire, les technologies numériques et les impératifs écologiques ne trouvent pas de réponse satisfaisante dans les modes actuels de financement. Ceux-ci peinent à assurer le fonctionnement courant et les investissements d'entretien. Les retards s'accumulent alors que le personnel est de plus en plus désemparé par les plans successifs d'économie. L'hôpital est un bien commun apprécié des Français, qui donne du sens à la solidarité et à l'engagement de l'État pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Les défis auxquels il est confronté doivent être résolus par un nouvel engagement national. Mieux inséré dans les parcours de soins, doté de capacités suffisantes pour rester à la pointe de la recherche et de l'innovation, garant de l'accès égal et de la participation des usagers à ses services, notre hôpital a un bel avenir devant lui ; nous devons lui en donner les outils. Or la fixation à 2 % de l'ONDAM hospitalier, même abondé de la hausse du forfait journalier, pose un nouveau cadre financier très contraint ; l'heure d'un nouveau « plan Hôpital » est donc venue, madame la ministre. Si l'on revient aux priorités, appréciables, de la stratégie nationale de santé, force est de constater qu'il n'est pas toujours aisé de les retrouver dans ce texte. La prévention est l'objet de mesures de fiscalité et d'une obligation concernant les vaccins ; l'Assemblée nationale y a ajouté le financement d'une consultation de dépistage pour les jeunes femmes. Nous approuvons la décision concernant les vaccins, tout en prêtant une grande attention au message envoyé par plusieurs sociétés savantes, dont le Collège national des généralistes enseignants, qui nous alertent sur les risques que l'obligation accroisse le phénomène de défiance, tant il est vrai que, en santé publique,

pilotée par le professeur Alain Fischer, qui insistait sur l'importance de plusieurs mesures : écoute de la population et des professionnels, transparence de l'information et des experts, diffusion d'informations validées, implication de l'école, campagnes de sensibilisation dans les médias ou encore facilitation de la pratique de la vaccination. de la pratique de la vaccination. C'est en complément de ces actions que le comité recommandait l'élargissement des obligations vaccinales de l'enfant. Il recommandait également la prise en charge à 100 % des vaccins obligatoires. C'est l'ensemble de ces axes qu'il faut appliquer pour réussir. Une politique de prévention en santé doit s'attaquer aux causes : au tabac, certes, mais aussi à l'alcool, aux polluants, dont ceux de l'air, et aux substances chimiques, notamment aux perturbateurs endocriniens, dont le rôle dans l'accroissement de nombreuses pathologies se révèle, au fil des études scientifiques, bien plus important que ce que l'on imaginait. imaginait. Que vienne le temps où la loi s'appuiera sur des recettes prélevées sur les polluants de l'alimentation pour financer un fonds alimentation-santé ainsi qu'une politique plus active en la matière ! À l'aune des évolutions sanitaires et sociales,

Nous approuvons cette volonté, mais il faudra mieux en préciser les objectifs : la lutte contre les inégalités, la prévention et la participation des usagers sont essentielles et les modes d'organisation doivent se penser Madame la ministre, votre projet contient des pistes intéressantes, mais aussi des ambiguïtés, relatives par exemple au tiers payant intégral, et il ne faudrait pas que cette ambiguïté se mue en un rendez-vous manqué avec la réduction des inégalités sociales. C'est un objet précieux, car il s'agit de la sécurité sociale et, au fond, pour ce qui concerne la santé, de la capacité de notre pays à réaliser de nouveaux progrès. Madame la ministre, ne nous décevez pas, portez la santé publique,

certains choix du Gouvernement présentés dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale recueillent l'approbation de notre groupe politique, que ce soit en matière de santé publique- c'est le cas de la lutte contre le tabagisme et de l'obligation vaccinale -ou en matière de politique de santé, avec le déploiement de la télémédecine et la mise en place d'organisations innovantes favorisant les initiatives des professionnels de santé. En revanche, nous ne vous suivrons pas pour ce qui concerne les retraités et les familles. Le basculement des cotisations salariales vers la CSG est présenté comme une mesure de « justice sociale [ ...] avec l'objectif d'une contribution équitable de l'ensemble des Français au financement de la protection sociale ». Mais où est la justice sociale ? En réalité, la mesure constitue une perte sèche pour huit millions de retraités qui avaient déjà subi une série de mesures sous les gouvernements précédents- la fiscalisation de la majoration de retraite pour charges de famille et la suppression de la demi-part des ces deux mesures ayant eu pour conséquence d'assujettir certains retraités au taux normal de CSG de 6,6 % et non plus au taux réduit de 3,8 % -, sans oublier le gel de leurs pensions depuis trois ans. Par ailleurs, alors que le versement des cotisations obligatoires ouvre toujours des droits, vous transférez sur la CSG des retraités les cotisations des actifs pour les indemnités de chômage. De cette façon, vous faites le choix de ne plus financer uniquement l'UNEDIC par les cotisations des salariés. Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons la proposition de nos rapporteurs de supprimer la hausse de 1,7 point de la CSG pour les retraités. Nous regrettons également que vous ayez fait le choix de continuer la politique familiale du gouvernement précédent. Nous estimons que cette politique doit être universelle, car elle est la preuve que l'État reconnaît le rôle fondamental de la famille dans la société, indépendamment de toute considération financière. Il est essentiel de comprendre que la vocation de la politique familiale n'est pas l'assistance, mais l'équité. Or la réduction du quotient familial et la modulation des allocations ont fortement fragilisé cette politique. Ce PLFSS prévoit une nouvelle baisse d'une des prestations familiales les familles seront progressivement concernées par la baisse du montant de la PAJE, certaines perdront leurs droits et d'autres verront le montant de leur prestation divisé par deux. Nous voterons donc la suppression de l'article 26 proposée par notre collègue Élisabeth Doineau. J'en viens maintenant au domaine médico-social. Je tiens à remercier notre rapporteur pour ce secteur, Bernard Bonne, qui nous a expliqué qu'une hausse tendancielle du niveau de l'ONDAM médico-social, bien que réjouissante, ne pouvait être un motif suffisant de satisfaction. du manque de places dans les établissements, dont les élus et les représentants associatifs se font les infatigables relais, je souhaite appeler votre attention sur deux sujets particuliers, dont l'urgence requiert qu'une réponse leur soit apportée lieu, je veux évoquer le cas de nos concitoyens atteints de handicap et contraints de recourir à des prises en charge à l'étranger. Voilà plus de deux ans que les alertes ont été déclenchées, notamment ici, au Sénat. Nous avons rendu des travaux, des préconisations ont été faites, mais peu de chose a été accompli. Des efforts ont, certes, été fournis, et je veux saluer les deux principales initiatives que constituent la « réponse accompagnée pour tous » et le fonds d'amorçage de 15 millions d'euros. Toutefois, l'ampleur et la cruauté du phénomène réclament des réponses d'une bien plus grande envergure 15 millions d'euros seulement pour contrer cet « exil des sans-solution » dont le coût s'élève à près de 400 millions d'euros ? Notre longue histoire de terre d'accueil nous inspire très justement l'horreur des départs contraints. Prompts à dénoncer ce mal quand il accable d'autres peuples, qu'attendons-nous pour y répondre quand il touche nos propres concitoyens ? L'intention du fonds d'amorçage doit être considérablement renforcée et, surtout, les conseils départementaux doivent être associés à la démarche. lieu, il n'y a pas que le secours financier qui soit salutaire. J'évoquais la « réponse accompagnée pour tous », la confection sur mesure d'un parcours personnalisé pour chaque personne handicapée. Oui, c'est la voie qu'il nous faut désormais emprunter. Oui, c'est aux structures et aux intervenants médico-sociaux de s'adapter aux besoins spécifiques de la personne. Mais à qui ce nécessaire et ambitieux projet est-il échu, sans qu'aucun moyen supplémentaire soit venu l'accompagner ? Aux maisons départementales des personnes handicapées, On veut en faire des interfaces performantes et réactives entre les publics touchés par le handicap et les acteurs chargés de leur prise en charge. Très bien ! Mais il faut alors leur donner les moyens d'assumer cette immense tâche. J'entends bien que les MDPH ont récemment été déchargées de missions qui excédaient leur coeur de métier, et c'est fort bien. Mais, là aussi, le pas franchi est trop timide. Nos MDPH sont trop souvent dépassées par l'ampleur des missions qui leur sont confiées,

La parole est à Mme Laurence Rossignol. Madame Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il est toujours un peu difficile de trouver la bonne distance à l'égard de sujets dont on a eu la responsabilité, entre une entre une indifférence qui serait totalement contrainte et la nécessaire liberté qu'il faut laisser à un ministre et à son gouvernement. Je veux évoquer devant vous deux sujets que je trouve importants, les modes

Les raisons en sont multiples, malgré les investissements réalisés et les choix budgétaires opérés, particulièrement par la CNAF, puisque, si ma mémoire est bonne, entre 2013 et 2016, 400 millions d'euros ont été consacrés à l'aide à l'investissement

hésitant à s'engager durablement dans la création d'établissements d'accueil de jeunes enfants. Sur ce sujet, ma conclusion, madame la ministre, est la suivante : je crois que nous sommes arrivés au moment où notre pays doit

que deux enfants meurent probablement chaque jour de violences à leur encontre ? Qui sait que 10 % des enfants sont victimes de violences sexuelles ? Qui sait que 80 % de ces violences ont lieu dans la sphère familiale ? ? La visibilité sur les violences faites aux enfants est infiniment moins grande, probablement parce que le déni est encore plus lourd, le tabou plus difficile à lever, la famille étant tellement présupposée être un lieu de protection et d'épanouissement qu'il est parfois fort difficile d'admettre qu'elle est aussi, pour les enfants, le premier lieu de violence et de maltraitance. J'en veux pour preuve que l'on en est au cinquième plan de lutte contre les violences faites aux femmes et seulement au premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Cela dit bien le décalage dans le temps entre les deux prises de

Madame la ministre, je sais que vous connaissez toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Je vous ai saisie récemment du cas particulier d'un adolescent atteint d'une forme rare de cancer, qui, malgré la qualité de la recherche en France, ne peut être traitée actuellement qu'aux États-Unis. J'ai obtenu auprès de vos services un accueil et une compréhension qui vous font honneur. Je vous remercie de votre engagement dans ce domaine. La question déborde d'ailleurs les cancers pédiatriques, puisque, dans ce cas, il s'agit d'une forme de cancer dont peuvent également être atteints des adultes. Le code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge forfaitaire de telles maladies. Il s'agit la plupart du temps de traitements coûteux. Il est heureux que notre législation ait prévu une telle possibilité de prise en charge. Je salue d'ailleurs l'engagement, dans ce domaine, des caisses de sécurité sociale, des médecins-conseils et des personnels, qui traitent ces cas avec beaucoup d'humanité. Je vous ai entendue vous engager à donner les moyens nécessaires à la recherche. Bien entendu, je vous fais confiance. Il faudrait que la recherche contre le cancer fasse partie des priorités de ce quinquennat, au même titre que certains axes prioritaires, que je ne conteste pas. Je suis convaincue qu'un effort peut être fait. Nous sommes tous prêts à apporter notre pierre à l'édifice, mais, en premier lieu, je souhaiterais que soient mis à contribution ceux qui produisent les médicaments. Certains médicaments sont plus rentables que d'autres, mais, aujourd'hui encore, certains marchés moins rentables sont insuffisamment investis par la recherche. C'est le cas des médicaments spécifiques aux traitements des cancers pédiatriques. Je souhaiterais qu'une contribution spéciale soit demandée à tous les fabricants de produits pour les traitements médicaux, pour les traitements de confort ou pour la cosmétique, que cette contribution soit partagée par moitié entre le fabricant et les consommateurs, le fabricant ayant ainsi la possibilité d'augmenter ou non le prix de vente de son produit de la moitié de la somme qu'il devra reverser pour la recherche, que cette contribution soit consacrée à la recherche contre le cancer, avec l'obligation d'en réserver la moitié au moins à la recherche spécifique contre les cancers pédiatriques. Je vous présenterai un amendement à ce sujet. Au reste, des associations de parents désemparés se sont créées pour recueillir des fonds privés afin de pouvoir faire face, dans l'urgence, à l'accompagnement de ces enfants. Ces parents, dans l'angoisse de ne pas pouvoir procurer à leur enfant les soins qu'il pourrait recevoir à l'étranger, créent des associations dans le but de pouvoir lever rapidement les fonds nécessaires au traitement de leur enfant. Il serait souhaitable que ces associations puissent bénéficier du statut d'intérêt général et, en conséquence, qu'elles puissent délivrer un rescrit fiscal aux donateurs, ce qui leur permettrait de lever beaucoup plus rapidement les fonds nécessaires. Bien entendu, tous les justificatifs devront être fournis, mais avec une priorité d'examen pour une réponse rapide, car dans ces cas dramatiques, on parle en jours ... Je veux maintenant intervenir sur les sujets de préoccupation principaux des Français de l'étranger tout d'abord, sur les « certificats de vie », question récurrente depuis des années, qui peine à trouver une solution. Nos compatriotes retraités résidant à l'étranger doivent prouver chaque année qu'ils sont vivants pour percevoir leur retraite. Quoi de plus normal ? beaucoup de nos compatriotes retraités résidant à l'étranger vivent loin d'une administration locale qui acceptera de justifier de leur existence. J'ai eu à traiter plusieurs cas de Français demeurant loin d'une représentation officielle qui puisse justifier de leur état. Pour s'y rendre, il faudrait qu'ils prennent l'avion ou le bateau et qu'ils en aient les moyens. Ceux qui sont trop âgés, malades ou sans ressources ne peuvent pas prendre ce risque. Par ailleurs, si le certificat n'est pas rédigé dans la langue du pays, qui voudra certifier ? J'ai même vu plusieurs cas de retraités venus passer quelques mois avec leur famille en France, ne pouvaient pas obtenir de la commune dans laquelle ils résidaient provisoirement auprès de leur famille ce fameux « droit à vivre dans la dignité » qu'est le certificat de vie. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, avec l'accord du Gouvernement, l'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, aux termes duquel « les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France peuvent envoyer aux caisses de retraite leurs certificats d'existence par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. » Ce dispositif devait entrer en vigueur le 1 janvier 2018. Le Conseil constitutionnel l'a déclaré contraire à la Constitution pour de simples raisons de procédure, considérant qu'il s'agissait d'un « cavalier législatif quelles solutions très pratiques et concrètes votre ministère peut-il apporter dans cet univers kafkaïen ? Un autre sujet concerne la situation de nos compatriotes expatriés qui rentrent en France, quelle qu'en soit la raison, mais bien souvent à la suite de la rupture de leur contrat de travail ou d'un problème familial, avoir la plupart du temps travaillé dans des entreprises de droit local qui ne les ont pas affiliés au régime de sécurité sociale français. Le bénéfice de la protection maladie universelle est subordonné à la justification d'une activité professionnelle ou à une résidence stable et régulière ininterrompue depuis plus de trois mois. des Français de l'étranger, la CFE, se retrouvent à leur arrivée en France et pour trois mois au moins sans assurance maladie, ce qui entraîne pour eux et pour leur famille des conséquences parfois gravissimes. Il serait souhaitable qu'ils puissent, dès qu'ils ont connaissance de leur retour en France, signaler cette situation auprès du consulat afin de pouvoir bénéficier d'une couverture sociale dès leur arrivée. Permettez-moi d'évoquer également la réforme du régime de la Caisse des Français de l'étranger. Cette réforme est en discussion depuis des mois, tant au niveau du conseil d'administration et de la direction de la CFE que dans un dialogue constant avec la direction de la sécurité sociale et votre cabinet. La réforme prévoit de nombreuses mesures, notamment une réflexion sur une prise en compte accrue de la composante liée à l'âge, une offre spéciale pour les jeunes de moins de 30 ans, une offre 100 % digitale, un « produit France » pour prendre en charge uniquement les soins en France, un objectif de remboursement clarifié pour les hospitalisations, etc. Il s'agit d'une réforme ambitieuse, qui doit se traduire par une nouvelle loi. Pouvons-nous espérer, madame la ministre, que ce texte puisse venir en discussion sans trop tarder ? tarder ? Pour terminer, j'évoquerai le problème crucial de la CSG-CRDS, qui inquiète nos compatriotes retraités. L'augmentation des prélèvements les préoccupe, car il en résultera une diminution de leur pouvoir d'achat, sans parler de leur assujettissement à ces prélèvements.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de l'ensemble de vos contributions. Je note déjà avec satisfaction que, sur un certain nombre de

Au total, sur les 7 millions de retraités qui connaîtront une augmentation de la CSG, 3,8 millions seront compensés, voire plus que compensés- ils gagneront en pouvoir d'achat par la suppression de la taxe d'habitation. J'ajoute que le PLFSS comportera des dispositions à destination des plus modestes, notamment la revalorisation du minimum vieillesse, qui augmentera dès le 1 avril 2018. Prenant en compte la politique fiscale et sociale dans son ensemble, nous sommes attentifs à l'équilibre d'ensemble des réformes, dont il est très important de retracer

qui assure une contribution de toutes les ressources productives. Il s'agit également d'une ressource adaptée au caractère de plus en plus universel de certaines branches, notamment

Sur la question de la dette et des besoins de financement de l'ACOSS, qui a été évoquée par beaucoup d'entre vous, le plafond de trésorerie de l'ACOSS devrait être porté à 38 milliards d'euros en 2018, contre 33 milliards d'euros Le montant de l'encours de dette de l'ACOSS ne pose pas de problème de financement dès lors que les taux à court terme demeurent bas, ce qui sera visiblement le cas en 2018, eu égard à la politique conduite par la Banque centrale européenne.

Nous prenons acte d'un changement de tarification des EHPAD, que nous allons accompagner, mais il ne s'agit évidemment pas là de l'ultime réforme de l'accompagnement de la perte d'autonomie de nos aînés, puisque nous savons que le nombre de personnes âgées dépendantes va tripler d'ici à 2050.

Monsieur Savary, vous avez évoqué la situation des retraites. Le Gouvernement est évidemment très attentif aux équilibres de la branche retraite à court et moyen termes. Nous allons suivre de très près les travaux du Conseil d'orientation des retraites, dont nous attendons le nouveau rapport.

Nous avons d'ores et déjà intégré dans nos hypothèses de travail une prévision d'évolution à court terme plus réaliste que celle qu'avait retenue le PLFSS pour 2017, mais nous nous adapterons au fur et à mesure.

le Fonds de solidarité vieillesse, il n'est pas exact de dire que la hausse du minimum vieillesse n'est pas financée. Je vous fais remarquer que le déficit du Fonds de solidarité vieillesse devrait diminuer- vous l'avez d'ailleurs relevé -de 200 millions d'euros en 2018.

devra tenir compte de toutes les sensibilités représentées au sein de cette assemblée, mais également de toutes les parties prenantes. La réflexion ne fait que commencer. On ne peut donc réduire le PLFSS

à une période où l'industrie pharmaceutique présentait un médicament ayant une indication. On a vu qu'avec une nouvelle politique visant à obtenir une première indication, souvent dans une niche, puis à développer progressivement de très nombreuses indications, le système des ATU ne permettait pas, une fois l'AMM octroyée, d'avoir accès

couverture vaccinale et sont, de ce fait, particulièrement sensibles aux épidémies. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une couverture vaccinale large pour éviter des décès d'enfants.

J'ai regretté, madame Cohen, que vous évoquiez le suicide d'un praticien à Grenoble. Si la qualité de vie des professionnels de santé

de la recherche et à accueillir toutes les populations, sans reste à charge. Nous allons travailler l'an prochain avec l'ensemble des acteurs pour que l'hôpital public retrouve la place qu'il n'aurait jamais dû cesser d'avoir.

sa cible de vue, à savoir l'accessibilité pour ceux qui en ont vraiment besoin, le plus rapidement possible. S'agissant du tabac, beaucoup de choses ont été dites sur les zones frontalières. Nous sommes parfaitement conscients de ce problème avec Gérald Darmanin. C'est la raison pour laquelle nous menons une politique acharnée de lutte contre la fraude

du commissaire européen à la santé, résolus à avancer vers une harmonisation de la fiscalité sur le tabac en Europe, avec la nécessité d'en faire réellement une priorité